En 1977, année durant laquelle Jacques Chirac devient maire de Paris, il est adjoint au maire et questeur de l’Hôtel de Ville. Au mois de septembre de la même année, il fait son entrée au Sénat, en même temps que Charles Pasqua. Roger Romani rejoint le groupe du Rassemblement pour la République (RPR) et devient membre de la commission des lois, avant d’être membre de la commission des finances. Il sera tout au long de sa vie politique un ardent défenseur du bicamérisme.

De 1993 à 1995, Roger Romani est ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, puis, de 1995 à 1997, ministre des relations avec le Parlement dans le gouvernement d’Alain Juppé.

dans la terre de Corse si chère à son cœur. C’est avec la même émotion que nous avons appris le décès de notre ancien collègue Jean Pierre Cantegrit. Devenu sénateur des Français de l’étranger, en 1977, Jean Pierre Cantegrit sera un pionnier en matière de protection sociale des Français expatriés. La loi du 17 juin 1980, sur le fondement de deux propositions de loi qu’il avait déposées au Sénat, étend la protection sociale aux Français de l’étranger non salariés, pensionnés ou retraités. En 1984, s’appuyant sur sa proposition de loi, un projet de loi prévoyant l’extension de la couverture à l’ensemble des citoyens français résidant hors de France sur la base d’une adhésion volontaire est adopté. Le texte instaure également la création d’une caisse autonome de sécurité sociale,

Merci

des affaires étrangères. Monsieur le ministre, mes chers collègues, l’Europe est à un tournant critique de son histoire. Cette nuit,

De l’autre côté de l’Atlantique, l’ancien président intérimaire Dimitri Medvedev indiquait ce matin que la Russie devait infliger une défaite « maximale » à l’Ukraine. C’est sans doute ce que Trump appelle « donner des signaux forts de paix ». La vérité, mes chers collègues, c’est que Poutine ne s’arrêtera pas à l’Ukraine, pas plus qu’il ne s’est arrêté à la Crimée en 2014. La nécessité de bâtir une défense européenne pour assurer la sécurité du continent doit donc maintenant être une évidence pour tous. Dans la douleur, tous les Européens en prennent conscience. La France défend depuis toujours l’autonomie stratégique européenne. Ursula von der Leyen a dévoilé des propositions d’ampleur, pour une montée en puissance militaire en urgence : 800 milliards d’euros pour permettre à l’Union européenne de s’équiper et de se préparer à la poursuite de conflits de haute intensité.

Avec l’abandon de l’aide américaine, les Européens devront fournir des efforts encore plus importants que par le passé. Pour se défendre, les États membres doivent se réarmer. Les domaines prioritaires sont identifiés : défense antiaérienne, missiles, artillerie, drones et antidrones. Monsieur le ministre, ma question est très simple comment pouvons nous accélérer enfin pour aider efficacement l’Ukraine et pour que notre base industrielle de défense soit le socle de la défense européenne ? Très concrètement, quelle est la position que vous défendrez demain ?

approvisionnements militaires en provenance des États Unis et d’ailleurs. Nous avons vécu pendant des décennies dans l’insouciance, acceptant progressivement que, dans

les sénateurs, depuis huit ans, sous l’impulsion du Président de la République, sous l’autorité du ministre des armées, vous avez adopté deux lois de programmation militaire nous permettant de revenir à un niveau qui se rapproche des 2 % du PIB et de réarmer notre pays. Il faut évidemment aller beaucoup plus loin. C’est tout l’objet du Conseil européen extraordinaire qui se tiendra demain. Ce sera l’occasion l’occasion de réaffirmer avec beaucoup de force que nous soutiendrons la résistance ukrainienne, qui est la première ligne de défense de l’Union européenne, et de nous accorder sur des moyens extraordinaires pour réarmer les pays européens. La présidente de la Commission européenne a fait une proposition : 800 milliards d’euros mis à disposition des États membres pour se réarmer. Cela passe à la fois par un assouplissement des critères du pacte de stabilité et de croissance, par une nouvelle facilité pour que les pays européens puissent s’endetter jusqu’à hauteur de 150 milliards d’euros, par une repriorisation

en train de se rallier. et Social Européen. Ma question s’adresse à M. le Premier ministre. Près de 64 % de nos concitoyens sont inquiets de l’évolution de la situation géopolitique depuis l’arrivée de l’administration Trump au pouvoir. On les comprend. La loi du plus fort redevient l’épine dorsale de l’ordre international, d’un côté, sous la pression de l’impérialisme russe, de l’autre, par la monétisation de la valeur paix par Washington. Monsieur le Premier ministre, vous avez tenu hier au Sénat des propos graves et responsables sur le changement brutal de la diplomatique américaine et ses conséquences sur le dossier ukrainien. Au nom du RDSE, j’ai pour ma part rappelé notre souhait de voir maintenue l’aide française et européenne à l’Ukraine. Nous le devons aux Ukrainiens, qui se sacrifient depuis trois ans, mais c’est nécessaire aussi pour garantir notre propre sécurité. J’ai également souligné combien la mise en œuvre d’une défense européenne crédible et concrète ne pouvait plus attendre. Nous serons attentifs aux conclusions du sommet européen

mêmes postures, les mêmes renoncements de la part des extrêmes. On sait où cela nous a menés : à l’impréparation de notre pays et à sa capitulation face aux nazis. Pour autant, nous ne pouvons pas seulement promettre à nos concitoyens, en particulier aux jeunes, une économie de guerre Il faut donner des signes d’espoir et d’apaisement. Le Président de la République s’adressera ce soir aux Français qui attendent des réponses. Monsieur le Premier ministre, aujourd’hui, quels sont les moyens et les atouts de la France et de l’Union européenne pour forcer la place du monde libre ? Bravo ! La parole

Les Français comme les autres Européens découvrent en cet instant, dans les jours que nous vivons, à quel point la situation est profondément déstabilisée.

américain prévoit que les équipements militaires ou les armes acquis auprès des États Unis ne peuvent pas être déclenchés s’il y a un veto des États Unis.

depuis le général de Gaulle jusque dans les huit dernières années, a défendu sans cesse l’idée que l’armement des Européens devait être un armement européen,…

de réarmement, de remise à niveau et de retour de l’indépendance dont nous avons besoin sera enfin comprise. Merci de l’avoir rappelé au Sénat. La parole est à Mme Audrey Bélim, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Je remercie également l’ensemble des élus locaux, des agents publics, mais aussi ceux du secteur privé et du secteur associatif, ainsi que les citoyens mobilisés depuis samedi, qui contribuent sans relâche, jour après jour pour, à ce que notre île se relève. Avec le dérèglement climatique, les cyclones s’intensifient Belal l’an dernier, Chido, Garance. Météo France indique que ses modèles robustes confirment que ceux ci seront de plus en plus forts dans l’océan Indien. En a t on tiré toutes les conséquences en termes d’adaptation ? Voilà un an, après Belal, j’alertais déjà sur la nécessité d’amplifier l’enfouissement du réseau électrique. À quoi sert d’élaguer les branches, quand les arbres se couchent désormais chaque année sur les fils ? 30 000 foyers sont toujours sans électricité ce matin. Je remercie les équipes. Reste qu’il faudra que les 25 % du réseau de basse et moyenne tensions encore aériens fassent l’objet d’une réflexion si l’enfouissement n’est pas possible. du réseau d’eau ? Après Belal, le préfet a demandé aux fournisseurs d’eau de s’équiper de groupes électrogènes en cas de besoin. Ce n’est toujours pas le cas partout. Comment cela est il possible dans une île où les dates de la saison cyclonique sont, hélas ! bien connues ?

Monsieur le ministre d’État, je vous remercie d’avoir lancé la procédure de catastrophe naturelle. Pour aller plus loin, pouvez vous vous engager à ce que le prochain Ciom (comité interministériel des outre mer) permette de parfaire et d’anticiper les actions en amont, durant et après ces événements, mais aussi nos stratégies à court, moyen et long termes ? Il y va de la protection de nos populations je vous remercie

devant ces cinq vies, cinq vies emportées par ce cyclone, cinq vies de trop. Je m’associe à vos condoléances et réaffirme notre soutien aux familles des victimes, ainsi qu’à l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais.

L’alimentation électrique a par ailleurs un impact sur l’eau potable. Elle doit être sécurisée. C’est pourquoi je souhaite que soit lancée une démarche de résilience de l’approvisionnement en eau pour faire face à la gestion des crises climatiques.

échec d’une vision obsolète, celle d’un monde régenté par les États Unis avec une Europe à leur remorque. Malgré tout, votre adhésion à un atlantisme sous domination américaine perdure. Le Gouvernement approuve t il le plan von der Leyen ? d’un tournant d’économie de guerre et de rationnement, à 800 milliards d’euros, c’est à dire d’une Europe politique de la défense, qui achète encore et toujours des armes américaines. Acceptons nous que nos armées soient placées sous le commandement d’un général américain obéissant à Trump ou songeons nous enfin à sortir de l’Otan ? Ce soir, devant les Français, le Président de la République fera t il le choix de l’escalade militaire ou celui d’un calendrier de la paix et de la sécurité collective ?

l’escalade, ce n’est pas celle des Européens ou des Ukrainiens. L’escalade, c’est celle de la Russie ! N’ayons aucune indulgence aucune indulgence vis à vis de Vladimir Poutine, aucune : assassinat d’opposants politiques, déportation des enfants ukrainiens, crimes de guerre, asphyxie de sa propre économie et de son propre peuple,… Vous avez trente ans de retard ! … pilonnage des pays européens de désinformation. Monsieur Savoldelli, est ce que les Européens déportent les enfants de la Russie ? Est ce que les Européens provoquent constamment, par une rhétorique nucléaire, la Russie de Vladimir Poutine ? L’agresseur dans cette affaire,

ont mis du temps avant de se rallier à cette idée là, mais tous ont pris pleinement conscience que les dépendances que nous avons accumulées vis à vis des États Unis, que ce soit dans le domaine de l’armement comme dans d’autres secteurs, sont tout à fait inacceptables et compromettent notre indépendance.

dans le monde qui vient, nous puissions défendre nos intérêts et notre vision du monde, laquelle, contrairement à celle de Vladimir Poutine, repose sur le droit international et la justice. Nous ne parviendrons à imposer nos intérêts et notre vision du monde qu’en étant plus forts et plus et plus indépendants. Quant à la sortie de l’Otan, ce n’est ni notre politique ni notre objectif. Voilà ! Au moins, c’est clair ! Notre objectif, c’est de nous emparer de l’Otan et, au moment où les États Unis s’en désengagent, d’y développer nos capacités, notre stratégie et notre vision pour, en Européens, assurer notre propre sécurité.

Il faut faire de la politique et assumer le débat démocratique. Que se passe t il aujourd’hui ? Les marchés applaudissent. Les profits s’envolent. Les commandes d’armes sont assurées par l’endettement public. Les Français ne veulent pas de la guerre. Exactement ! Personne ne veut de la guerre

Il faut sortir du duo Trump Poutine ! Les Ukrainiens n’auront ni la paix ni la souveraineté et notre sécurité ne sera pas plus garantie. Le monde a changé, il est multipolaire. Il faut être aux côtés des Ukrainiens et des Européens

a annulé l’autorisation environnementale de l’A69, qui doit relier Castres à Toulouse, au motif que la « raison impérative d’intérêt public majeur » n’était pas prouvée. Pour les Tarnais, que je représente avec mon collègue Philippe Folliot, c’est un véritable séisme et un immense désastre. Le chantier s’arrête à moins de dix mois de la mise en service : 70 % des ouvrages d’art sont réalisés et plus de 300 millions d’euros ont été dépensés ! C’est un désastre social pour les 1 000 ouvriers qui se sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain. C’est un désastre économique pour les entreprises. C’est un désastre écologique et paysager pour les habitants. C’est une cicatrice de 53 kilomètres – et les compensations environnementales ne seront jamais mises en place. C’est un désastre politique, enfin, pour tous les élus, et un désastre financier pour l’État et le contribuable. À court terme, que va devenir ce chantier ? Nous vous remercions d’avoir immédiatement annoncé faire appel du jugement et demandé un sursis à exécution, mais quelles sont les chances de reprise du chantier, et avec quel calendrier ? À plus long terme, ce jugement pourrait faire jurisprudence. C’est une véritable épée de Damoclès qui est désormais suspendue au dessus de tous les futurs projets d’infrastructures, petits et grands. N’y a t il pas urgence à faire évoluer la loi pour éviter que notre pays ne se retrouve définitivement sous cloche ? La

En tant que ministre de la République, je respecte pleinement l’État de droit. Mais respecter l’État de droit, ce n’est pas se résigner à l’insensé et à la situation des 1 000 personnes qui, comme vous l’avez dit, madame la sénatrice, madame la sénatrice, se retrouvent sans travail du jour au lendemain. C’est aussi avoir le courage de dire quand une situation devient absurde. L’A69 est un projet porté par un territoire tout entier, qui se bat depuis trois décennies pour son désenclavement. La région Occitanie, le département du Tarn, les collectivités locales et les entreprises l’attendent désespérément. Comment ne pas être stupéfait ? Comment comprendre qu’un projet déclaré d’utilité publique, ayant fait l’objet de six recours déjà rejetés, dont les autorisations environnementales avaient été validées et dont les travaux sont avancés à 70 %, comme vous l’avez dit, puisse se retrouver brutalement à l’arrêt Face à cette situation, bien sûr que l’État fera appel ! Nous demanderons rapidement un sursis à exécution. Notre détermination est intacte : les travaux doivent reprendre au plus vite. Mais cette situation révèle, vous l’avez dit également, un mal profond, l’empilement des procédures, qui paralyse notre action publique. Ce qui arrive à l’A69 aujourd’hui menace tous nos projets de demain, qu’il s’agisse de sécuriser vos routes ou de moderniser vos réseaux ferroviaires. Le droit environnemental est essentiel, sauf quand il devient un instrument d’obstruction systématique. C’est pourquoi

La parole est à M. Grégory Blanc, pour le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.

Après l’annonce de fermeture, d’une brutalité inouïe, la seule chose que l’entreprise dit à ses salariés, aujourd’hui, c’est : « Continuez de produire à cadences soutenues ! Mais vous aurez à peine plus qu’à La Roche sur Yon, il y a six ans, avant les bénéfices records, avant le choc d’inflation. Michelin vient de réaliser, en 2024, un résultat opérationnel de 3,4 milliards d’euros. Et ce groupe refuse de lâcher quelques millions d’euros pour reconnaître le travail d’une vie, assurer, malgré le licenciement, que la maison sera bien payée. En français, cela porte un nom : bien plus que du mépris, c’est de la maltraitance ! Madame la ministre, il y aurait bien des questions à vous poser sur l’échec des politiques industrielles du Gouvernement. Les syndicats de Michelin alertent déjà sur la situation à Montceau les Mines et à Troyes.

l’annonce du départ de Michelin de Cholet, dans votre département, a été un choc, comme à Vannes. Ce fut un choc pour les salariés, pour leurs familles et pour ces villes tout entières. La priorité du Gouvernement est bien celle de la loi : la continuité professionnelle et salariale

comme elle l’a fait par le passé. Le Gouvernement s’active aussi pour aider à la recherche d’un repreneur : c’est le rôle du réseau des commissaires aux restructurations économiques. Nous travaillons avec le cabinet qui a été mandaté par Michelin et les administrations centrales pour faciliter l’identification de ces repreneurs. Plus largement, France Travail se tient aux côtés des

Madame la ministre, quand Michelin délocalise les machines, c’est illégal. Comment comptez vous faire respecter la loi ? En 2024 encore, c’est à dire il y a quelques semaines, Michelin faisait alterner dans ses usines temps de travail à plein régime et chômage partiel. C’est nous tous qui payons le chômage partiel… En 2024, Michelin touchait encore des aides à l’emploi. Je demande que le Gouvernement agisse. Les 1 200 familles de Cholet et de Vannes vous regardent. Pour qu’un gouvernement dure, il faut aussi poser des actes

Ma question, monsieur le ministre, est d’un autre ordre. N’avez vous pas le sentiment que ce qui se passe en Ukraine est le révélateur de la fin d’un système international fondé en 1945 sur deux valeurs, la démocratie et la liberté ? La parole est à M. le ministre de l’Europe et des affaires étrangères.

le Premier ministre l’a rappelé à la tribune du Sénat comme il l’avait fait à la tribune de l’Assemblée nationale –, nous assistons au réveil des logiques d’empires qui, ne reconnaissant pas les frontières, foulent aux pieds l’ordre international fondé sur le droit que nous avons contribué à bâtir sur les ruines de la Deuxième Guerre mondiale.

que l’ONU a été fondée pour écarter le risque de la guerre, sur le principe simple du respect de l’intangibilité des frontières. Nous voyons ces logiques d’empires se déployer sous différentes formes ici et là, et nous retrouvons dans les déclarations de la nouvelle administration américaine les germes de cet impérialisme que l’ONU avait réussi à contenir. alors ? Soyons clairs : dans un moment comme celui ci, nous pouvons nous détourner de cet héritage, de cette construction dont nous sommes les dépositaires, considérant que, à notre tour, nous devons entrer dans ces logiques d’empire. Mais nous ne le ferons pas, car nous considérons que seuls le droit et la justice peuvent garantir à la communauté internationale une paix durable. Les logiques d’empires, dans lesquels certains voudraient nous entraîner, nous mèneraient un jour ou l’autre dans des guerres que nous n’aurons pas choisies. Mais pour défendre nos intérêts, les intérêts de la France et notre vision du monde qui repose sur le droit international et la justice, nous n’aurons pas d’autre choix que d’être beaucoup plus forts et beaucoup plus indépendants.

à l’échelle internationale, et nous n’aurons plus voix au chapitre. C’est pourquoi le moment que nous vivons est si important. En renforçant l’Europe et en renforçant la France, nous avons l’occasion,

Monsieur le ministre, je n’avais pas l’intention de vous entraîner dans une logique d’empire… En revanche, je m’interroge sur le fonctionnement de l’ONU, vous savez, cette organisation qui est censée assurer la paix dans le monde.

Sinon, cela ira de mal en pis. Puis, très clairement, l’Europe et l’Occident doivent se réarmer moralement, militairement, pour être en état de faire face. La France, notamment, a un rôle éminent à jouer. Ne nous laissons pas engluer dans des organisations internationales qui ne jouent plus le leur

et indépendants. Ma question s’adresse à M. le ministre d’État, ministre des outre mer. Permettez moi tout d’abord d’avoir une pensée pour nos amis de la Réunion, après le passage du cyclone Garance, qui a fait cinq morts, de nombreux blessés et d’importants dégâts.

Il y a trois semaines, les agents du syndicat mixte de gestion de l’eau et de l’assainissement de Guadeloupe ont entamé une grève, qui s’est poursuivie par un conflit autour du paiement des jours de grève. Ces actions ont touché l’ensemble des communes de la Guadeloupe et privé d’eau la moitié de la population au plus fort de la crise. En plus des conséquences humaines et sanitaires, l’effet est dramatique pour l’économie locale. L’eau est indispensable à de nombreux secteurs d’activité

du droit de grève est légitime, il est inacceptable de prendre en otage les habitants en les privant d’accès à l’eau. Je salue le travail des collectivités territoriales de Guadeloupe, qui poursuivent les investissements destinés à fiabiliser et moderniser les infrastructures de production et de distribution d’eau potable. Au delà du seul cas de la Guadeloupe, d’autres territoires ultramarins font également face à des difficultés de gouvernance, des manques en capacités techniques et des fragilités financières, qui impactent la qualité et la continuité du service public de l’eau. Le comité interministériel des outre mer (Ciom) tenu en juillet 2023 avait acté Monsieur le ministre d’État, où en sommes nous, et quelle est votre feuille de route sur le sujet ? Le dossier de l’accès à l’eau est prioritaire et devra être central lors du prochain Ciom. Il n’est plus possible que, en 2025, sur le territoire de la République, nos concitoyens n’aient pas un accès continu à

Je condamne fermement ces méthodes irresponsables. Les auteurs de ces actes de malveillance doivent être identifiés et poursuivis par la justice. Je salue les agents non grévistes qui ont relancé les sites de production grâce à la sécurisation assurée par les forces de l’ordre. Ce syndicat mixte fait l’objet d’un contrat d’accompagnement renforcé depuis 2023. L’État se tient à ses côtés en apportant un soutien financier et technique.

sur lequel nous pouvons nous retrouver et sur lequel nous devons être intransigeants, c’est la sécurité de nos compatriotes. Je suis ministre de l’intérieur et la sécurité est ma priorité.

43 % de ceux qui sont retenus dans les CRA sont de nationalité algérienne. Ils sont libérés au bout de 90 jours. Que faire si nous n’obtenons pas de laissez passer consulaires

On veut le faire taire ? Eh bien, je vous le dis, nous, nous ne nous tairons pas Merci, monsieur le ministre. La sécurité, c’est ce que l’État nous doit, c’est ce qu’il doit à chaque citoyen français. Je crois que chacun en est convaincu ici. Vous démontrez aussi que vous en êtes convaincu et que vous savez comment renforcer la sécurité des Français. Puissiez vous en convaincre le Président de la République comme vous en avez convaincu le Gouvernement !

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Georges Berthoin, à qui l’histoire offrit un destin européen aux côtés de Jean Monnet, et que je voulais évoquer en ces heures sombres, fut associé à la rédaction du traité créant la Communauté européenne de défense (CED), une sorte de plan Schuman élargi. Il reconnut ultérieurement qu’il était heureux que ce projet n’ait pas abouti en l’état, car, si le volet militaire était prêt – et l’on parlait tout de même d’une armée intégrée de plus de 500 000 hommes –, il n’en allait pas de même du volet politique. Je crains, monsieur le ministre, que ce ne soit aujourd’hui l’inverse. Les conclusions du sommet de Londres et celles du Conseil européen qui se tiendra demain à Bruxelles devraient acter l’existence d’une volonté politique servie par des organes – ceux de l’Union européenne et de l’Otan – susceptibles de donner corps au projet d’une défense européenne. Reste néanmoins le volet militaire.

Faute de disposer des chaînes de montage et des personnels nécessaires – car doubler le budget des armées sans augmenter leurs ressources humaines n’aurait aucun sens – auprès de qui l’Union européenne va t elle acheter les matériels nécessaires dans les mois à venir ? À Israël, à la Turquie ou à la Corée du Sud ? La

! Le Sénat se bat pour contrecarrer une logique planificatrice et dirigiste imposée par les gouvernements successifs. Voilà quatre ans que nous essayons de concilier la sobriété foncière avec un vrai accompagnement des élus.

à son compte la consommation foncière qui en résulte. L’État se dit aux côtés des maires, mais ne fait rien pour que les préfets tiennent compte de la loi votée au Parlement. Les exemples sont nombreux… L’État prétend territorialiser, mais il entend maintenir une date couperet en 2034 pour l’application du ZAN à toutes les communes. L’État veut davantage de logements sociaux,

je vous remercie de votre question. Nous avons déjà eu l’occasion d’échanger et nous allons continuer à tracer notre chemin ensemble, si vous en êtes d’accord. Dès la semaine prochaine d’ailleurs, nous aurons l’occasion d’échanger lors de l’examen de cette proposition de loi, déposée par vous même et le sénateur Cambier.

Depuis, un projet de révision de l’arrêté tarifaire nous alerte. Il pénaliserait de nombreuses initiatives locales citoyennes œuvrant de longue date, en cohérence avec leur localisation, en faveur de la promotion des énergies renouvelables, en particulier Même si je comprends la nécessité de réduire la dépense publique, ce changement abrupt de cap heurte de plein fouet des initiatives vertueuses, la lisibilité des règles, ainsi que la stabilité des modèles économiques.

indispensable à la réussite de la décarbonation de l’énergie dans les territoires, risque d’aggraver notre retard, mais également d’exposer le pays à des sanctions financières à l’échelon européen. Madame la ministre, une telle décision n’entre t elle pas directement en contradiction avec nos objectifs nationaux de décarbonation ? En conséquence, allez vous revenir dessus ? dessus ? La parole est à Mme la ministre déléguée chargée du commerce, de l’artisanat, des petites et moyennes entreprises et de l’économie sociale et solidaire.

Ma question s’adresse à M. le ministre d’État, ministre des outre mer. Cinq personnes ont perdu la vie après le passage du cyclone Garance. J’adresse ici tout mon soutien et celui de mon groupe à leurs familles. Des centaines de familles réunionnaises sont sinistrées ; je souhaite leur exprimer ma solidarité. Je tiens également à saluer l’action de nos élus, de nos pompiers, de nos soignants et des agents des services publics ou privés ainsi que de l’État, qui sont venus en aide à l’ensemble de la population dans ces circonstances tragiques. Après la dévastation de l’archipel mahorais, c’est La Réunion qui a été à son tour durement éprouvée ce 28 février, avec des vents dévastateurs de plus de 200 kilomètres heure et des pluies diluviennes. Avec la chute de 21 pylônes de très haute tension, cette catastrophe majeure a privé des familles de toit et a endommagé de nombreuses habitations. À l’heure actuelle, 40 000 foyers sont sans électricité, et 30 000 sont privés d’eau. Des pans entiers de l’économie locale sont touchés ; des commerces, des entreprises et des bâtiments publics sont fortement endommagés. Nos agriculteurs voient leur production totalement détruite, alors qu’ils se relevaient à peine du cyclone Belal de 2024, pour lequel les aides tardent à être versées. (CHU) a été inondé, ce qui complique considérablement la prise en charge des patients, alors même que les risques sanitaires post cycloniques sont connus et peuvent entraîner des épidémies.

pour venir en aide aux familles réunionnaises sinistrées, pour alléger les charges de nos entreprises et pour accompagner nos collectivités, dont les budgets sont déjà contraints ? Allez vous préconiser des dispositifs concrets de prévention des risques face aux phénomènes climatiques,

ministre d’État, ministre des outre mer. Madame la sénatrice Malet, vous avez eu raison de rappeler la mobilisation de tous. Depuis la levée de l’alerte rouge samedi matin, les services de l’État et les collectivités sont pleinement mobilisés pour venir en aide à la population, réparer les premiers dégâts et rétablir la situation. Les effectifs engagés sont particulièrement importants. Ainsi, 900 personnels des forces de sécurité

Je me rends dès ce soir à La Réunion, afin d’être aux côtés de la population éprouvée, des élus locaux et de l’ensemble des équipes de secours. Nous ferons un état des lieux précis des actions prioritaires pour soutenir les habitants sinistrés de l’île et permettre la reconstruction.

de compléter ces annonces au regard de ce que je pourrais constater avec l’ensemble des professionnels. J’espère que nous pourrons répondre le plus vite possible aux attentes – elles sont fortes – de nos compatriotes réunionnais.

Deux semaines plus tôt, dans le quartier Saint Chamand, il y avait eu un homme abattu et cinq blessés graves. C’est une mécanique implacable qui broie des vies ! Comment ne pas penser au capitaine de police Éric Masson, assassiné en pleine ville sur un point de ? Trois ans après, la situation a empiré. La violence et les deuils se multiplient. Les habitants vivent sous tension. La peur paralyse. Aujourd’hui, les transports en commun sont bloqués dans tous ces quartiers. La délinquance est là, s’affirme et s’étale.

vous avez intégré Avignon au dispositif Villes de sécurité renforcée, comme Grenoble, Rennes et d’autres. Je veux ici saluer cette décision. Il faut tirer les leçons des échecs passés. Votre prédécesseur, Gérald Darmanin, enchaînait des opérations spectaculaires pour faire « place nette ». Mais une place nette sans projet, c’est une place vide, qui devient perdue pour notre République ! Saint Chamand, Monclar, La Rocade… Dix ans de violence ! Combien de services publics, de centres sociaux et d’associations laissés à l’abandon ? Quand on abandonne un quartier, il se remplit d’autres lois que celles de notre République. Il faut un État qui protège, une police formée et dotée de moyens réels, une justice efficace et juste. Je veux ici saluer le travail du préfet Thierry Suquet celui des forces de l’ordre et des acteurs de terrain emmenés par la maire Cécile Helle, qui, avec des moyens contraints, tentent de ralentir une telle spirale. Quels moyens durables et pérennes comptez vous mettre en place pour Avignon ? Les criminels, eux, n’attendent pas ! Monsieur le ministre d’État,

et le système de notation censé indiquer la qualité nutritionnelle des aliments. Or ce système est contesté. Défavorable aux produits traditionnels, tels que les fromages au lait cru et la charcuterie, il soulève de nombreuses craintes chez les producteurs et les filières de qualité, qui en dénoncent les critères. En 2020, la Commission européenne envisageait de rendre le Nutri score obligatoire à l’échelle de l’Union européenne. Cependant, le 28 février 2025, un vote de la Commission européenne a validé le retrait du Nutri score obligatoire ; à cette occasion, la France s’est abstenue. Cet abandon répond à des préoccupations légitimes. Je les avais déjà soulevées avec d’autres ici auprès de vos prédécesseurs en insistant sur la nécessité d’éviter une obligation qui aurait fragilisé les filières de qualité.

comme pour le comté chez moi, ou pour toutes les magnifiques salaisons françaises, c’est que le classement de ces produits remarquables était très mauvais. Ils

L’arrêté est à ma signature. Je ne l’ai pas encore signé. Je ne sais pas quelles sont mes marges de manœuvre pour corriger les effets négatifs, mais croyez bien que je m’y intéresse de très près. Cela étant,

de politique énergétique sont pour le moins sinueuses, pour ne pas dire branchées sur courant alternatif. La dernière déclaration du Président de la République, avec la fameuse formule !, laissait

locales photovoltaïques avec des installations intégrées à des bâtiments, c’est à dire sans dénaturer les sols naturels. C’est précisément le cas du secteur dit S21. Des installations photovoltaïques de moins de 500 kilowatts sur des bâtiments sont déjà financées par des collectivités locales, des particuliers, voire des exploitants agricoles. Or les professionnels de la filière que nous avons rencontrés nous disent que nous ne sommes pas à l’abri d’un nouveau court circuit général. En effet, le décret que le Gouvernement s’apprêterait à prendre signerait

aujourd’hui, le coût des installations du photovoltaïque sur toiture est deux fois plus élevé que celui du photovoltaïque au sol

orienté vers des installations plus performantes et économiquement viables de plus grande puissance. Encore une fois, l’électricité ne se stocke pas et il n’est pas du tout vertueux de produire de l’électricité l’on ne peut pas consommer. Dans ce cadre, un arrêté spécifique sur le photovoltaïque au sol plus compétitif sera publié avant la fin du premier trimestre de 2025, afin d’encourager ce type d’installations et de diversifier les sources de production d’énergies

Madame la ministre, il y a des contrats qui ne sont pas encore signés, mais qui sont déjà bien engagés. Les collectivités comme les particuliers ont pris des engagements sur la base d’aides publiques actées précédemment. Ce qui est reproché par les acteurs de la filière, c’est la brutalité de la baisse annoncée. Ils ne sont pas hostiles à un changement des règles du jeu, mais pas comme cela.

visant à lutter contre la vie chère en renforçant le droit de la concurrence et de la régulation économique outre mer, présentée par M. Victorin Lurel et plusieurs de ses collègues Conformément à l’article 74 de la Constitution ainsi qu’aux articles L.O. 6213 3, L.O. 6313 3 et L.O. 6413 3 du code général des collectivités territoriales, le Sénat a consulté les conseils territoriaux de Saint Barthélemy, de Saint Martin et de Saint Pierre et Miquelon ainsi que l’assemblée territoriale de Wallis et Futuna sur cette proposition de loi. Dans sa délibération du 24 février 2025, le conseil territorial de Saint Pierre et Miquelon a émis un avis favorable sur ce texte.

Invention des injonctions structurelles, réglementation des marchés de gros, interdiction des accords d’exclusivité d’importation et de distribution, renforcement des pouvoirs de l’Autorité de la concurrence, décrets sur les carburants, création du bouclier qualité prix (BQP) : nous avons alors agi vite et, je crois, puissamment.

Nous sommes aujourd’hui en 2025 et, disons le, les structures de marché n’ont que trop peu évolué. L’opacité perdure, les rentes persistent, les concentrations et les dominations demeurent, l’activisme et l’ingéniosité sont toujours à l’œuvre pour contourner les lois. Avec cette proposition de loi,

Convaincu que de petits pas constituent souvent de grandes avancées, je pense que ce texte est équilibré et qu’il pourrait recueillir l’agrément de notre assemblée. Toutefois, compte tenu de la prégnance du fléau de la vie chère et de la complexité des structures de marché, qui, hélas ! comme le dit le ministre,

Ces amendements tendent à prévoir des mesures fortes afin d’encadrer et de plafonner les marges arrière, de sécuriser les commerçants locaux face aux oligopoles qui contournent la loi de 2012,

qui, en quelques semaines, a eu l’audace de placer la lutte contre la vie chère parmi ses priorités. Il est d’ailleurs intéressant de noter que notre débat a lieu quelques jours après l’entrée en vigueur de l’exemption de TVA

d’agir en faveur du pouvoir d’achat – on y refuse, pour le moment, de baisser l’octroi de mer. Monsieur le ministre, vos mots sont forts, vos engagements sont fermes. Une volonté nouvelle semble avoir été affirmée. Elle doit dès aujourd’hui se traduire en actes. Ne décevez pas l’espoir suscité. Vous voulez, vous pouvez, vous devez donc agir ! Au delà des lois, de nombreuses mesures réglementaires peuvent d’ores et déjà être prises

remisés dans les tiroirs et soumis à la critique rongeuse des souris… Nous espérons que cette proposition de loi prospérera ; à partir de ce soir, je n’en suis plus propriétaire. Monsieur le ministre, toutes les idées sont sur la table, toutes les bonnes volontés s’expriment et nos peuples attendent des mesures fortes. Faites vôtres les avancées conquises aujourd’hui. Je suis intimement convaincu que la discussion de ce texte peut utilement donner matière à une nouvelle grande loi contre la vie chère, qui serait soutenue par le Gouvernement. Je suis prêt à vous aider et à alimenter la

de toutes nos forces. Je comprends désormais toutes ces mobilisations récurrentes contre la vie chère dans ces territoires. Je remercie l’auteur de la proposition de loi,

beaucoup de produits étrangers doivent d’abord entrer sur le territoire métropolitain avant d’être réexpédiés vers les outre mer, et ce afin de respecter les normes sanitaires et réglementaires.

en raison de l’étroitesse des marchés, la plupart des entreprises locales souffrent d’un manque de débouchés, ce qui les empêche très souvent de réaliser des économies d’échelle. Leur compétitivité prix est d’autant plus faible qu’elles subissent la rigidité des coûts du travail.

en vue de les contraindre à déposer les comptes de leur société. Je vous présenterai un amendement visant à préciser les modalités de cette astreinte. Les compromis trouvés à l’article 2

Selon moi, le réel problème réside moins dans la transmission de documents par les entreprises que dans la communication entre les services de l’État d’informations déjà détenues. À cela s’ajoute la complexité de la structuration juridique et financière des grandes sociétés intégrées verticalement ou en situation d’oligopole transversal sur le commerce. Ces deux phénomènes nuisent à la transparence et à la compréhension de la structure des marges. Dans les faits, ces groupes mutualisent leurs coûts d’approche, conservent tous les gains et les économies d’échelle, maîtrisent les coûts de financement et du foncier, ce qui empêche l’émergence d’autres opérateurs. Pour toutes ces raisons, nous devons reconnaître que ces grands groupes sont des passages obligés.

Mes chers collègues, je resterai mobilisée sur les enjeux de la vie chère dans les outre mer. La commission des affaires économiques continuera d’apporter son soutien critique et vigilant à toute mesure permettant d’améliorer structurellement la situation. C’est dans cet esprit que nous avons examiné les amendements déposés sur ce texte. Je terminerai mon propos par une remarque d’ordre plus général. Monsieur le ministre, les territoires d’outre mer ont véritablement besoin de vous pour réaliser une transformation en profondeur de leur économie, et ce sur plusieurs volets. améliorer la concurrence – ce texte y contribue déjà – ; réduire les rigidités des marchés ; renforcer les structures de financement et de paiement des petites entreprises pour améliorer leur rentabilité et réduire leur besoin en fonds de roulement concentrer les efforts d’investissement sur la modernisation des ports et des plateformes logistiques, ainsi que sur la transition énergétique et l’autonomie alimentaire, afin de développer l’agriculture locale ; œuvrer à l’intégration régionale de ces territoires.

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, madame le rapporteur, monsieur l’auteur de la proposition de loi, mesdames, messieurs les sénateurs L’histoire des outre mer dans la République est celle d’une longue marche vers l’égalité, vers l’égalité réelle. » Ces mots ne sont pas les miens,

il m’est malheureusement impossible d’affirmer que cette marche vers l’égalité est terminée. Mais je peux dire en revanche que Victorin Lurel, avec d’autres bien sûr, avancer en la matière. La loi dont je viens de parler a constitué un tournant dans l’encadrement des pratiques commerciales ultramarines.

insupportable et insoutenable pour nos compatriotes ultramarins. Cela constitue une véritable fracture sociale, qui nourrit un sentiment d’inégalité et un ressenti d’injustice. Ces derniers s’aggravent dangereusement.

un plan de bataille complet, structurel, sérieux, crédible, qui s’attaque méthodiquement à tous les facteurs qui concourent à la cherté de la vie dans les outre mer. Ce plan se résume en cinq mots. Le premier mot est : « concurrence Je tiens depuis plusieurs semaines un propos de vérité, qu’il aurait fallu sans doute tenir depuis bien longtemps. Oui, le partage et la chaîne de valeur outre mer ne sont pas

Pour mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles, je ne crois pas en la seule bonne volonté des acteurs. Je veux remettre en première ligne de ce combat l’Autorité de la concurrence, renforcer ses moyens et la rapprocher du terrain. Sinon, cela ne marchera pas. Je souhaite avancer sur la création en son sein d’un service d’instruction spécialisé et consacré aux outre mer. En outre, nous le savons, il faudra également renforcer les moyens et les équipes de la DGCCRF.

deuxième mot est : « transparence ». Trop d’entreprises ne se conforment pas à leur obligation de publication des comptes. Je suis déterminé à renforcer les sanctions et à les rendre plus dissuasives. L’article 1 constitue

point. De son côté, l’État a avancé. La promulgation de la loi de finances nous a permis de tenir notre engagement d’appliquer une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité. Il nous reste à imaginer un mécanisme pour

copier coller d’autres rapports et qu’elles nous fourniront des éléments précis pour nous permettre d’agir. Les distributeurs, enfin, ont déjà réalisé un effort sur leurs marges, mais les marges arrière fortement à l’opacité sur la formation des prix des produits et sur la réalité des bénéfices réalisés par les grands groupes. Je souhaite donc, comme vous, renforcer la transparence sur ce sujet.

Pour sortir d’une économie de comptoir, il faut rompre avec la dépendance aux importations, favoriser la production locale et l’autonomie alimentaire.

Les idées sont nombreuses sur ce sujet. Je pense bien sûr aux deux propositions de loi que nous examinons aujourd’hui. À cet égard, je remercie le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et son président Patrick Kanner d’avoir choisi de consacrer sa niche parlementaire entière aux outre mer, plus particulièrement à la problématique de la vie chère. Je le reconnais bien là

faudra faire converger toutes ces initiatives et vous pouvez compter sur ma totale détermination et sur une très grande clarté de ma part. Je sais que je suis attendu sur les actes plus que sur les discours. Il y a bien sûr ce qui relève d’une réalité économique l’éloignement qui augmente les coûts, l’étroitesse des marchés qui empêche les économies d’échelle et, parfois, la faiblesse des infrastructures. Mais il y a aussi ce qui relève de la tromperie,

que l’on peut constater ici en France hexagonale ; dans les territoires ultramarins qui connaissent une double insularité, ce phénomène est encore plus grave. La vie chère dans les outre mer

50 % de plus – ou les communications – jusqu’à 35 %. Le panier alimentaire hexagonal moyen coûte par exemple 46 % plus cher à La Réunion. Ces chiffres, qui traduisent des écarts avec l’Hexagone pour le moins criants, sont d’autant plus importants qu’ils sont à considérer à l’aune d’un niveau de pauvreté tout aussi alarmant. Je rappelle que le niveau hexagonal se situe à 15 %. La vie chère en outre mer est donc une réalité, une réalité profondément injuste.

un effet négatif sur les prix auprès des consommateurs : étroitesse des marchés, éloignement géographique, nécessité d’importer depuis l’Europe, possibilités limitées de productions locales et existence de certains oligopoles

pense par exemple à la possibilité récemment octroyée à plusieurs collectivités ultramarines de déroger au marquage CE afin de pouvoir importer des produits de construction issus de pays de leur zone géographique. C’est une mesure de bon sens.

qui ont notamment pour mission d’analyser les prix, les marges et leurs évolutions. Je pense aussi aux outils issus de la loi de 2012 relative à la régulation économique outre mer, dont notre collègue Victorin Lurel était notamment permis d’instaurer un bouclier qualité prix sur des produits essentiels et de renforcer la transparence sur les prix, notamment dans le secteur de la grande distribution. C’est d’ailleurs, entre autres, sur l’une des mesures de cette loi que la présente vise à revenir. Dans sa version initiale, le texte prévoyait de transformer l’obligation, pour certaines entreprises, de transmettre leur comptabilité analytique sur demande en une transmission systématique annuelle. Si nous comprenons bien l’objectif de cette mesure, qui est de renforcer la transparence des entreprises et des prix, nous partageons toutefois le point de vue de Mme le rapporteur : cette mesure serait bien trop lourde pour les entreprises, elle pourrait même être dissuasive pour l’implantation de nouvelles d’autant plus que l’obligation existante de dépôt annuel des comptes est déjà trop peu respectée. Nous soutenons donc la version de la commission qui vise à renforcer les sanctions en cas de non respect des obligations existantes et qui crée la possibilité pour le préfet de demander au tribunal de prononcer une injonction avec sanction d’astreinte dans le cas où les comptes n’auraient pas été transmis. L’objectif n’est donc autre que de contraindre davantage au respect du droit existant. Les outils existent, mais ils doivent être appliqués. La lutte contre la vie chère, pour être efficace, nécessite aussi, je le pense, un projet plus global,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je tiens tout d’abord à remercier mon collègue Victorin Lurel et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain d’avoir permis, par l’inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat,

Cette réalité pèse lourdement sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens ultramarins et alimente des mobilisations récurrentes. Ce texte apporte certaines avancées, en renforçant la régulation économique et en stimulant la concurrence, deux leviers essentiels pour briser les situations de monopole ou d’oligopole qui maintiennent artificiellement des prix élevés dans de nombreux secteurs. Mais comment garantir une véritable concurrence, si les marchandises peinent à arriver à destination ou si les coûts logistiques deviennent insoutenables ? À Saint Martin, le problème de la vie chère est aggravé par la double insularité et un modèle économique qui repose essentiellement sur l’importation. Chaque hausse des coûts logistiques se traduit immédiatement par une augmentation des prix dans les commerces. Avec la suppression de certaines dessertes maritimes directes, Saint Martin devient encore plus dépendante des plateformes portuaires régionales pour son approvisionnement. Cela signifie plus de transbordements, de délais et de surcoûts. Nos commerçants et entrepreneurs, déjà confrontés à une concurrence complexe avec la partie néerlandaise de l’île, risquent de voir leur situation se détériorer encore davantage. Les consommateurs, eux, paient le prix fort sans disposer

Les commerçants locaux subissent de plein fouet l’instabilité des livraisons. Un conteneur retardé, c’est tout un stock qui manque en rayon, obligeant les détaillants à passer par des circuits plus coûteux.

Face à ces défis, nous devons sortir d’une dépendance excessive aux routes d’importation traditionnelles et mieux intégrer nos territoires aux circuits économiques de la Caraïbe. Cela passe par une meilleure coopération avec les îles voisines, qui pourraient devenir des plateformes logistiques stratégiques pour diversifier nos sources d’approvisionnement. Cela passe aussi par la levée des freins réglementaires qui compliquent les échanges avec nos voisins caribéens, alors que ces circuits pourraient être une solution efficace pour réduire les coûts et améliorer la fluidité des livraisons. Nous devons également renforcer notre partenariat avec les acteurs régionaux du commerce et du transport pour ne pas être uniquement tributaires des grandes compagnies maritimes, qui réorganisent leurs routes sans trop se soucier des réalités locales. Saint Martin, située au cœur de la Caraïbe, doit pouvoir tirer parti de sa position géographique en renforçant ses liens commerciaux avec les autres îles de la région. Nous ne pouvons plus nous permettre d’être des marchés captifs, entièrement dépendants de décisions prises à des milliers de kilomètres. Nous nous devons de rester lucides : les mécanismes de régulation économique ne pourront pas produire leurs effets si les coûts de transport continuent de croître sans contrôle. C’est pourquoi il m’apparaît nécessaire d’avoir un cadre de régulation du transport maritime adapté aux réalités ultramarines. Les grands armateurs réorganisent leurs lignes en fonction de leur rentabilité. C’est leur logique et elle est compréhensible. Mais qui veille à ce que ces réorganisations ne laissent pas nos territoires dans une situation encore plus précaire ? L’État doit également prendre ses responsabilités, en surveillant de près l’évolution des coûts du fret maritime afin d’éviter des hausses injustifiées qui viendraient aggraver le phénomène Enfin, il est vital que des solutions soient envisagées pour sécuriser l’acheminement des biens essentiels vers nos territoires, notamment en facilitant les connexions avec les ports voisins de la région. Il ne suffit pas d’adopter des textes sur la concurrence si, dans le même temps, nos territoires restent à la merci de décisions logistiques prises sans considération pour les réalités locales. Cette proposition de loi est une avancée et je la soutiens, mais elle ne suffira pas si nous ne prenons pas la mesure du problème logistique. Sans une logistique fiable, il n’y a ni concurrence ni baisse des prix. Nous devons donc faire en sorte que ce texte soit suivi de mesures concrètes pour garantir un accès stable et équitable aux biens de consommation en outre mer. Nous ne pouvons pas rester spectateurs des bouleversements en cours dans le transport maritime. Nos concitoyens ultramarins attendent des réponses. Il est de notre responsabilité d’anticiper ces défis et d’agir pour que la régulation économique en outre mer soit non pas un vœu pieux, mais une réalité tangible dans le quotidien des Ultramarins. La parole

nous voilà une fois de plus réunis pour débattre de la question de la vie chère dans nos territoires ultramarins, comme un écho qui revient incessamment, cette continuité historique et structurelle traversant les décennies, comme les océans.

À cette époque déjà, des rapports mettaient en lumière une concentration des acteurs économiques et des marges exorbitantes pratiquées par certains distributeurs. Le constat n’est donc pas nouveau sur l’étroitesse et la structure des marchés, les multiples contraintes insulaires, l’éclatement des chaînes d’approvisionnement menant à des situations oligopolistiques,

la loi Lurel de 2017 que les auteurs du présent texte entendent actualiser. Voilà quelques exemples d’outils législatifs mis en place face à une fissure sociale grandissante, pour ne pas dire béante. Nous tentons en somme de réguler les prix et les marges depuis de nombreuses années, de résoudre le problème dit de la vie chère, mais force est de constater que, malgré la juxtaposition et la multiplication de textes et de mesures aux effets parfois éphémères, vivre dignement reste un combat du quotidien en outre mer. Nous devons en tirer les leçons.

Mais restons lucides : ce texte, aussi utile puisse t il paraître, contient des mesures encore trop isolées qui, malheureusement, n’infléchiront pas seules le cours des choses. Agissons ensemble, mes chers collègues, monsieur le ministre ! Un sursaut est impératif, mais il doit être collectif. Le problème de la vie chère appelle une réponse globale et ne saurait être résolu par des initiatives isolées ou partielles. Ce dont nous avons besoin, c’est d’un engagement ferme et d’une vision renouvelée pour prendre à bras le corps ce sujet et en traiter tous les symptômes – vous en parliez à l’instant, monsieur le ministre. Cette thématique de la vie chère touche intimement la question du pouvoir d’achat et des modèles économiques. Ce sursaut doit passer par des mesures touchant à la régulation économique, aux moyens de l’Autorité de la concurrence, aux circuits d’approvisionnement, aux conditions de transport, aux frais d’approche, mais aussi à l’emploi, à la jeunesse, au foncier, au logement, à l’aménagement du territoire, à la fiscalité, à la transition énergétique ou encore aux infrastructures. Ce sursaut doit aussi passer par le dépassement d’une vision somme toute étriquée sur l’existence d’un outre mer uniforme et global ou au mieux binaire –

et nous formulerons le mois prochain des propositions pour agir contre ce fléau qui ne doit plus être une fatalité pour nos territoires. Ce combat – c’en est un ! – appellera des moyens à la hauteur, si nous partageons tous la même ambition. Nos territoires français des trois océans s’épuisent, las d’être chéris dans les discours, mais trop peu considérés dans les faits. Nous aurons besoin de vous, monsieur le ministre, et je sais que vous avez identifié ce sujet comme une priorité. La Polynésie française n’échappe pas à ces maux, elle les combat avec difficulté et avec les moyens dont elle dispose. J’appelle d’ailleurs l’État, au delà des questions statutaires, à accompagner notre collectivité sur ces questions qui pèsent sur les citoyens français que sont aussi les Polynésiens. Soyons vigilants, car cette précarité économique qui s’enracine alimente dans tous nos territoires un sentiment de désaffection à l’égard de l’État, qui apparaît tantôt impuissant tantôt insensible aux appels à l’aide des populations écrasées par le diktat des prix outre mer.

et à un engagement sincère pour considérer, enfin, dans toute sa mesure cette frustration qui croît. Il nous faut mobiliser l’État, nos collectivités et toutes les forces vives, avec l’engagement et l’intensité qu’appelle une cause de portée nationale dépassant les postures et les joutes politiciennes. Notre force réside dans notre capacité à agir ensemble. Ne laissons ni la vie chère ni les inégalités qui se creusent éroder ce lien précieux qui nous unit au sein de la République. Dans ce contexte,

Nous sommes réunis aujourd’hui, dans le cadre de la niche parlementaire du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, pour travailler sur deux propositions de loi relatives aux outre mer. Il s’agit d’une bonne nouvelle sur le papier, mais sur le papier seulement, car le timing est tout de même malheureux. Consacrer une niche exclusivement à des sujets ultramarins durant les jours gras, en plein carnaval, quand on connaît l’engouement pour ces festivités dans nos territoires ! Il fallait y penser… y penser… Certains de nos collègues évoquent le roi Vaval et le brûlent au soleil – je peux les comprendre. À Saint Pierre et Miquelon, nous l’appelons Bulot et il brûlera sur le quai sous la neige jonchant actuellement le sol de mon archipel. C’est aussi cela la richesse de nos outre mer J’ai néanmoins l’honneur d’être présent devant vous pour évoquer cette proposition de loi visant à renforcer le droit de la concurrence et de la régulation économique outre mer, texte intéressant pour lutter contre la vie chère dans nos territoires.

Les OPMR ont un rôle important à jouer sur le coût de la vie dans les territoires ultramarins. Ils sont capables d’apporter la concertation et la cohésion nécessaires.

Sur un territoire aussi maritime que le mien, tout changement dans ce domaine ne serait pas sans conséquence. Mesurer un changement de méthode d’approvisionnement d’un territoire, c’est comprendre son influence sur le coût de la vie et permettre la compréhension des difficultés de sa population. Mes chers collègues, je ne veux pas gâcher la fête, mais cette méthode essentielle de concertation ne peut pas partir en confettis et cet amendement ne doit pas finir sur le quai, réduit en cendres aux côtés du roi Bulot.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, imaginez un instant devoir payer 40 % plus cher votre panier de courses quotidien. C’est non pas une fiction, mais bien la réalité pour nos compatriotes ultramarins. Ce chiffre n’est pas nouveau. Il traverse les décennies, cristallise les colères, alimente les mobilisations. Je tiens tout d’abord à remercier notre collègue Victorin Lurel de cette proposition de loi, ainsi que notre rapporteure Évelyne Renaud Garabedian, dont le travail a permis d’améliorer le texte et d’atteindre un équilibre entre régulation et et compétitivité. Le constat est implacable : la vie chère en outre mer est une réalité. Les causes en sont multiples et bien identifiées. L’éloignement géographique impose des coûts logistiques importants, qu’il s’agisse du fret maritime ou aérien. La taille restreinte des marchés locaux limite les économies d’échelle et rend les importations plus onéreuses. À cela s’ajoute une taxe spécifique, l’octroi de mer, qui, bien que source essentielle de financement pour les collectivités, renchérit encore davantage les prix des produits de première nécessité. Ces facteurs cumulés font de la vie chère une réalité quotidienne de plus en plus insupportable pour nombre d’Ultramarins, dont les revenus, eux, ne suivent pas la même courbe ascendante. Cette situation économique a des conséquences sociales alarmantes. Les mobilisations contre la vie chère sont récurrentes, des Antilles à La Réunion, en passant par Mayotte. Depuis septembre dernier, la Martinique connaît une vague de contestation qui témoigne d’une exaspération profonde face à la cherté de la vie. Pour répondre à cette urgence, certains avancent une explication supplémentaire le manque de concurrence. Il est vrai que, dans plusieurs secteurs clés, comme la grande distribution, les carburants ou les télécommunications, quelques acteurs dominent le marché et bénéficient d’une position privilégiée. treize groupes d’entreprises contrôlaient plus de 50 % des marchés aux Antilles et en Guyane et réalisaient près de 18 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Ces structures, souvent familiales, sont accusées de verrouiller l’accès à de nouveaux entrants et peuvent conserver des marges importantes.

Il serait donc hasardeux d’en faire le seul ou principal facteur de la vie chère. L’un des axes majeurs du présent texte est le renforcement du contrôle des concentrations et des fusions. Il s’agit d’empêcher la constitution de monopoles ou d’oligopoles qui faussent le marché. Nous soutiendrons toujours ce qui peut favoriser les conditions d’une concurrence pure et parfaite. La commission a ainsi introduit des ajustements notables, comme l’abaissement du seuil de notification des fusions de 5 millions à 3 millions d’euros pour le commerce de détail ou encore l’élargissement des possibilités de saisine des différentes autorités. Ces avancées permettront une surveillance plus fine des pratiques commerciales et une meilleure régulation du marché. Cependant, réguler ne signifie pas entraver. Si la concentration des acteurs économiques pose problème en cas d’abus de position dominante, il ne faut pas pour autant faire des entreprises des boucs émissaires. Une approche punitive pourrait avoir des effets pervers : fuite des capitaux, exil des talents ultramarins, affaiblissement du tissu économique local. Or nos entreprises sont non pas des adversaires, mais des partenaires d’une économie plus juste et compétitive.

Aujourd’hui, 24 % des entreprises martiniquaises seulement déposent leurs comptes, contre 85 % dans l’Hexagone. Cette opacité empêche une régulation efficace et limite la capacité des autorités à identifier d’éventuels abus. La commission a ici apporté des modifications bienvenues : la transmission automatique a été remplacée par une procédure d’injonction, ce qui permet un contrôle plus ciblé et proportionné, assorti d’une sanction en cas de non transmission. En effet, veillons collectivement à ne pas faire preuve d’un excès bureaucratique. Chaque nouvelle obligation administrative représente des charges supplémentaires pour les entreprises, dont les coûts sont répercutés sur les consommateurs.

Bienvenue dans la République de la bureaucratie ! Cette accumulation de contraintes aurait asphyxié les acteurs économiques sans garantir une réelle efficacité. Rappelons nous, mes chers collègues, qu’en octobre dernier nous avons adopté, en première lecture, le projet de loi de simplification de la vie économique

aussi à nos entreprises ultramarines. Évitons une inflation réglementaire qui, sous couvert de transparence, risquerait de freiner l’investissement et la croissance. Chaque mot supplémentaire dans notre arsenal juridique est un euro en moins dans le portefeuille des Ultramarins. Enfin, la lutte contre la vie chère en outre mer ne peut être efficace sans une politique d’ensemble que notre délégation sénatoriale entend proposer dans son prochain rapport d’information sur la lutte contre la vie chère. La dépendance excessive aux importations est un frein au développement économique des territoires ultramarins. Encourager l’agriculture locale, développer les industries de transformation, investir dans des infrastructures logistiques modernes : tous ces leviers permettraient de réduire les coûts et d’assurer une plus grande autonomie économique. Lutter contre la vie chère en outre mer, c’est défendre un principe fondamental d’égalité économique et sociale. Le groupe Union Centriste votera ce texte. La lutte contre la vie chère en outre mer exige une politique cohérente, structurelle et durable. La parole

Entre survivre et vivre, le choix est vite fait. Nos peuples aspirent à une vie digne, ce qui implique la lutte contre la vie chère dans nos pays dits d’outre mer. Les peuples d’outre mer ont le droit de manger et boire au même prix que les Français de l’Hexagone, c’est une évidence. Mais vivre de nos terres, voilà notre vraie richesse. D’ordinaire, ces territoires sont traités dans les assemblées parlementaires au simple détour d’un article de loi autorisant le Gouvernement à légiférer par ordonnances. Cette proposition de loi

Ces territoires sont un terrain de jeu pour le développement d’un capital sans gêne ni scrupule qui outrepasse les règles, loin des contrôles qui se pratiquent dans l’Hexagone. Que ce soit en Kanaky, en Martinique, à La Réunion, en Guyane ou encore à Mayotte, les évènements récents ont mis en lumière ce que vivent nos peuples. Dire « non » à la vision coloniale de l’économie et « oui » à la dignité : voilà ce que les mobilisations, de la Martinique jusqu’aux rues de Paris, ont fait résonner. Cela souligne notre volonté indéfectible de défendre l’émancipation sociale et économique des nôtres.

C’est non pas l’éloignement de ces territoires qui est la source de la vie chère outre mer, mais un système et ses acteurs économiques hérités directement du colonialisme. Leurs marges abusives et leur manque de transparence n’en sont qu’un symptôme, enfin exposé dans le débat public hexagonal.

Fabien Gay en commission, avec la caution de l’État depuis des années. Nous regrettons que les modifications du texte initial amoindrissent la portée de ce texte. Nous avons la responsabilité, par de plus fortes mesures, de redonner espoir à nos peuples,

Mes pensées vont aux familles touchées, aux habitants confrontés aux dégâts considérables et à tous ceux qui, sur le terrain, œuvrent sans relâche pour protéger, secourir et reconstruire. Plus que jamais, la République doit se trouver au côté de La Réunion dans cette épreuve et apporter un soutien à la hauteur de ses besoins. L’outre mer est une composante essentielle de notre nation, une partie intégrante de notre identité républicaine. Ces territoires portent en eux la richesse de l’Histoire, la diversité des cultures, mais aussi une réalité sociale et économique qui exige de notre part une attention constante et des actions à la hauteur des enjeux. La République est une et indivisible, mais elle ne doit pas être uniforme. » Ces mots d’un ancien président du Sénat originaire de nos outre mer – Gaston Monnerville, pour ne pas le citer – nous rappellent la nécessité de prendre en compte les spécificités et les défis des territoires ultramarins dans la lutte contre les inégalités. Nous avons une responsabilité impérieuse : faire en sorte que nos compatriotes ultramarins ne soient pas condamnés à une vie marquée par l’injustice économique et les difficultés quotidiennes.

Les coûts excessifs des produits de première nécessité, des services essentiels et des biens de consommation courante exacerbent un sentiment d’abandon et d’inégalité, alimentant ainsi un profond malaise social. Ce malaise n’est pas nouveau. Il s’est exprimé avec force lors de grandes mobilisations sociales qui ont marqué ces dernières décennies. Qui pourrait oublier la grève générale de 2009 aux Antilles, lorsque des milliers de citoyens se sont levés contre la cherté de la vie et les inégalités criantes ? Qui pourrait ignorer les révoltes sociales récurrentes en Guyane ou à La Réunion, où les mêmes revendications refont surface avec une intensité grandissante ? Derrière ces colères, il y a des familles qui peinent à joindre les deux bouts, des travailleurs qui voient leur pouvoir d’achat s’effondrer, des jeunes qui n’entrevoient pas d’avenir digne dans leur propre territoire. Les chiffres parlent d’eux mêmes et sont accablants. Les écarts de prix entre la métropole et les départements et régions d’outre mer atteignent 10 % à 15 % en moyenne, avec des pics de 30 % à 40 % pour certains produits en Polynésie française et en Nouvelle Calédonie. Les produits alimentaires, qui représentent une part importante des dépenses des ménages, coûtent environ 30 % plus cher qu’en métropole. Cette réalité a des conséquences dramatiques : 900 000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté dans ces territoires. Plus d’un Ultramarin sur deux doit renoncer régulièrement à certaines dépenses du quotidien pour pouvoir se nourrir ou payer ses factures. Cette situation n’est pas tolérable. Face à cette injustice, les mesures ponctuelles ne suffisent plus. Nous devons agir en profondeur, avec une stratégie claire et une volonté politique affirmée. Des leviers existent : une meilleure régulation des circuits d’importation et de distribution, la lutte contre les monopoles, le renforcement des dispositifs de soutien au pouvoir d’achat, ainsi qu’un véritable plan de développement économique adapté aux spécificités ultramarines. Il est également essentiel d’encourager la production locale, de soutenir l’entrepreneuriat et de réduire la dépendance aux importations pour pour offrir des solutions de rechange durables et viables. Monsieur le ministre d’État, nous devons entendre le désespoir et la lassitude de nos compatriotes d’outre mer. Il est urgent de leur apporter des réponses concrètes et immédiates. La justice sociale et l’égalité territoriale doivent non pas rester de simples principes inscrits dans nos discours, mais devenir une réalité tangible pour celles et ceux qui souffrent au quotidien de ces inégalités. Nous avons le devoir de faire vivre la promesse républicaine sur l’ensemble du territoire national, sans distinction ni oubli. Les débats que nous avons aujourd’hui ne doivent pas déboucher sur un énième constat d’échec. Ils doivent être le point de départ d’un engagement renouvelé et d’une action ambitieuse en faveur des territoires ultramarins.

la vie chère en outre mer est non pas une fatalité, mais la conséquence de déséquilibres structurels qu’il nous revient de corriger. Aujourd’hui, nous consacrons le temps de la niche parlementaire du groupe socialiste à un enjeu essentiel : une économie plus juste pour nos concitoyens ultramarins. Depuis 2012, notre collègue Victorin Lurel porte avec constance cette cause. Ses lois de 2012 et 2017 ont marqué des avancées, mais certains dispositifs doivent être consolidés, pour mieux protéger les distributeurs locaux et garantir une concurrence équitable. Si le texte soumis à notre examen est resserré en trois articles, il constitue une avancée significative et un levier indispensable pour la suite. Il envoie un signal clair : les Ultramarins ne doivent plus être prisonniers d’un système économique inéquitable. Son objectif prioritaire est de renforcer la pression sur les entreprises qui ne respectent pas leur obligation légale de dépôt des comptes sociaux.

soient pleinement effectifs, notamment pour protéger les distributeurs locaux. Nous demandons ensuite que les conditions générales de vente établies au niveau national entre fournisseurs et distributeurs s’appliquent de manière transparente et non discriminatoire dans les outre mer. D’autres groupes parlementaires partagent cette exigence, et nous espérons parvenir à une rédaction mettant fin à ces distorsions de concurrence.

qui est perçue par le distributeur en contrepartie des services qui sont rendus à un fournisseur : la mise en avant de produits, la publicité sur les lieux de vente et les attributions d’emplacements privilégiés dans les magasins. Les marges arrière améliorent directement la rentabilité, mais, malheureusement, elles ne contribuent pas à la transparence. Contrairement aux remises et aux rabais commerciaux qui sont consentis par les fournisseurs, elles ne viennent pas en déduction du prix d’achat des produits. C’est une pratique qui est critiquée pour son impact négatif sur les prix à la consommation, certaines de ces marges arrière pouvant aller jusqu’à représenter 35 % du prix qui est facturé.

remercie, madame le rapporteur, de me laisser seul face à Victorin Lurel. Vous ne savez pas ce que c’est…

Le manque de transparence qui entoure cette pratique accentue la difficulté pour les fournisseurs, rend plus délicat le contrôle de l’État et empêche trop souvent, en pratique, que ces marges arrière soient répercutées sur le prix de vente aux consommateurs. Et c’est bien sur ce point que nous devons agir.

dire. En revanche, l’obligation d’inscription des avantages obtenus sur les factures d’achat va dans le bon sens et facilitera les contrôles réalisés par la DGCCRF. J’ai déjà eu l’occasion de le souligner, c’est avant tout en matière de transparence que nous devons avancer. Aussi,

les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles, notamment d’un accord exclusif d’importation prohibé par l’article L. 420 2 1 du code de commerce, peuvent déjà, comme le disait Mme le rapporteur, saisir le juge judiciaire afin d’obtenir réparation du préjudice subi.

De ce fait, même s’ils n’en sont que des substituts, leur impact concurrentiel les rend comparables, ce qui fragilise l’équilibre économique du territoire. C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’élargir la notion de concurrence, en y intégrant les produits comparables. Il vise ainsi à soutenir l’autonomie alimentaire des territoires ultramarins concernés, qui nous est chère à tous, en renforçant la compétitivité des produits locaux et en garantissant une concurrence équitable, qui passe par une protection efficace contre les pratiques commerciales déloyales.

L’article 2 de cette proposition de loi tend à limiter le renforcement de groupes déjà en position dominante sur les marchés ultramarins. C’est un objectif louable en vue d’accroître la concurrence localement. Cependant, les spécificités de chacun des territoires doivent être prises en compte. La densité commerciale, par exemple, n’est pas la même partout. Ainsi, en Guyane, où la population est en pleine croissance, il faut favoriser l’installation de grandes surfaces commerciales, car certaines parties du territoire en sont encore dépourvues. La population ne dispose que de petits commerces de proximité, dont on sait qu’ils proposent moins de produits, et à des prix plus élevés. Or la limitation que tend à instaurer cet article risque de ralentir, voire de bloquer le déploiement de ces commerces, faute de groupes aux dimensions suffisantes. Cet amendement vise donc à adapter l’article 2, pour tenir compte de ces réalités.

s’agissant du bouclier qualité prix. Si leur nécessité et leur importance ne sont pas à prouver, leurs moyens restent trop faibles. C’est pourquoi cet amendement vise à clarifier le statut des OPMR, afin qu’ils puissent disposer de leur pleine capacité opérationnelle et accomplir leurs missions, dans l’intérêt des consommateurs et des acteurs économiques locaux.

de doter ces structures de moyens leur permettant d’assurer leurs missions.

dans la difficulté, dans un territoire où le coût de la vie est déjà très élevé. Le dispositif est simple : permettre à l’observatoire des prix, des marges et des revenus d’être saisi, afin de rédiger une étude d’impact sur une décision de modification structurelle des conditions de la desserte maritime internationale du territoire. J’entends l’argument, qui me sera rétorqué, consistant à questionner la nécessité d’un avis conforme en bout de course. Cependant, je maintiendrai cette proposition, car elle est essentielle pour mon territoire et repose sur deux piliers : l’évaluation et la concertation. L’évaluation, tout d’abord : la desserte maritime en fret de Saint Pierre et Miquelon constitue la colonne vertébrale de toute l’activité économique et de toute la consommation de ce territoire isolé. Modifier la méthode d’approvisionnement peut entraîner des conséquences très négatives pour le coût de la vie. Une étude d’impact est donc nécessaire pour optimiser la prise de décision. La concertation, ensuite, puisque, comme vous le savez, mes chers collègues, les services de l’État, les élus et les forces économiques d’un territoire siègent au sein de l’observatoire des prix, des marges et des revenus. Ainsi, on ne laisse plus la place à l’arbitraire, le dialogue prime et les décisions sont réfléchies et incontestables.

du Nord. Aux relations et négociations souvent difficiles avec le voisin canadien, s’ajoute désormais la politique protectionniste et agressive de notre autre voisin, les États Unis de Donald Trump.

l’autorité administrative peut se charger de l’opération. Cette proposition me paraît positive. Elle permettra de mieux faire connaître l’ensemble des travaux et études que réalisent les OPMR. Ces observatoires devront donc réaliser chaque année un rapport annuel,

Écologiste et Républicain, de la proposition de loi expérimentant l’encadrement des loyers et améliorant l’habitat dans les outre mer, présentée par Mme Audrey Bélim et plusieurs de ses collègues

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez moi tout d’abord de rendre de nouveau hommage aux victimes réunionnaises, après le passage du cyclone Garance sur notre île. J’adresse, en votre nom à tous, nos pensées émues à leurs familles et à leurs proches.

Dans cette préface, Micheline Jacques écrivait : « Les bouleversements géopolitiques récents, les enjeux climatiques et écologiques de réduction de l’empreinte carbone font de la nécessité de disposer de référentiels propres aux outre mer une urgence, tant du point de vue des matériaux que des modes de construction.

Je souhaite remercier également la présidente de la commission des affaires économiques, Mme Dominique Estrosi Sassone, experte du logement, comme chacun le sait, qui a examiné avec un œil bienveillant ce travail des filières socioprofessionnelles ultramarines.

une conviction très simple : la République doit être partout chez elle, en Ardèche comme à La Réunion, dans les Alpes Maritimes comme en Martinique, en Essonne comme en Guyane.

80 % des foyers ultramarins sont éligibles au logement social. Pourtant, nombre d’entre eux n’ont d’autre choix que de se tourner massivement vers le parc locatif privé, tant la construction de logements, notamment sociaux, s’est effondrée ces dernières années. L’Association des communes et des collectivités d’outre mer (Accd’om) a distribué un questionnaire sur cette proposition de loi à l’ensemble des maires ultramarins. Le résultat est unanime : de Mayotte à la Guyane, en passant par la Guadeloupe, l’expérimentation dans les communes volontaires – j’insiste sur cet adjectif – est ardemment souhaitée. C’est à cette attente que le Sénat doit répondre aujourd’hui.

Nous devons être à la hauteur de ce vote historique, continuer à avancer et réaliser des progrès concrets sur ce sujet crucial dans notre hémicycle : la maison des territoires, c’est nous

car le surcoût lié à l’importation des matériaux pourrait être réduit en utilisant des ressources produites sur le territoire ou dans le bassin géographique. Il s’agit d’intervenir directement sur le coût des loyers, donc d’agir, une fois encore, sur le pouvoir d’achat, c’est à dire sur le pouvoir de vivre. qu’a tenus Manuel Valls à nos collègues députés, le 19 février dernier : « Pour réduire les prix, il nous faut rompre avec un modèle infantilisant, parfois ubuesque. Limitons les importations – très coûteuses – depuis l’Hexagone ou l’Union européenne à ce qui est strictement indispensable. Mayotte importe son bois de Lettonie,

Ce peut être le cas des normes australiennes, parfois plus protectrices en matière anticyclonique. Le passage du cyclone Garance à La Réunion nous montre que nous pouvons encore progresser en matière d’adaptation de nos constructions. L’Association des maires du département de La Réunion (AMDR) note que, dans l’est de l’île, 80 % des habitations ayant perdu leur toit datent de moins de quinze Ne pourrions nous pas nous inspirer de ce qui fonctionne ailleurs ? Pour amplifier les initiatives prises à Mayotte, tout en nous inspirant de la dynamique néo calédonienne, nous vous proposons de créer des comités relatifs aux produits de construction. des comités relatifs aux produits de construction. Ces comités seront chargés de contribuer à la nécessaire mise en œuvre de l’exemption de marquage CE, en tenant compte des besoins de la production, des spécificités et des contraintes locales.

Nous devrions permettre à la Guyane de s’inspirer de ces référentiels. Étant donné l’important travail mené par l’ensemble des acteurs publics et privés dans le cadre des Assises de la construction durable en outre mer, le dialogue et la concertation doivent présider à la rédaction des décrets d’application.

Ces sénateurs représentent l’ensemble des bassins océaniques et des groupes politiques comptant des élus ultramarins. Il faut conclure, ma chère collègue. L’adaptation des normes dans les outre mer est non plus une option, mais une nécessité. Elle permettra de créer des emplois locaux, de réduire notre empreinte carbone, de développer notre résilience face au changement climatique et de valoriser nos savoir faire traditionnels.

chers collègues, j’ai, moi aussi, une pensée particulière pour nos compatriotes réunionnais, frappés par le cyclone Garance la semaine dernière. Le bilan est lourd, trop lourd. Je sais, monsieur le ministre, que nous pouvons compter sur une action forte de l’État et des acteurs locaux pour venir en aide aux sinistrés le plus rapidement possible. J’en viens J’en viens à la proposition de loi de notre collègue Audrey Bélim, dont je sais l’engagement pour son territoire, particulièrement en ces moments difficiles. Ce texte vise à renforcer l’adaptation des normes en outre mer dans trois domaines

autour du logement abordable, en permettant aux collectivités d’outre mer qui le souhaitent de mettre en œuvre un dispositif d’encadrement des loyers. En effet, l’expérimentation actuelle d’encadrement des loyers, prévue par la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, les 48 communes bénéficiaires sont toutes situées dans l’Hexagone. À l’époque, aucune commune ultramarine n’entrait dans la catégorie des communes situées en zone tendue, éligibles au dispositif. Ce n’est plus le cas depuis que la liste des communes situées en zone tendue a été actualisée en août 2023. Or, à cette date, le délai fixé par la loi Élan pour candidater à l’expérimentation d’encadrement des loyers était déjà échu. La commission a donc estimé légitime de donner aux collectivités d’outre mer la possibilité de candidater à ce dispositif, comme ont pu le faire celles de l’Hexagone. s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la vie chère outre mer, même si le poste le plus emblématique en la matière reste l’alimentation, avec des écarts de prix pouvant s’élever jusqu’à 40 % entre l’Hexagone et la Guadeloupe, par exemple. Les loyers ne sont pas en reste : ils représentent une part très significative du budget des ménages, plus encore que dans l’Hexagone, compte tenu du moindre niveau de revenus de nos compatriotes ultramarins. Bien évidemment, l’encadrement des loyers est un outil qui doit demeurer facultatif et être laissé aux mains des élus locaux. Il ne doit pas nous conduire à ménager notre soutien à l’investissement locatif,

La commission a donc renforcé le dispositif proposé par notre collègue Bélim, sans pour autant interférer dans l’expérimentation actuelle d’encadrement des loyers en métropole, qui arrive à échéance à la La ministre du logement a diligenté une mission d’évaluation de cette expérimentation. Il est essentiel de ne pas la prolonger avant d’en avoir dressé le bilan. Nous avons ainsi créé une nouvelle expérimentation dans les collectivités ultramarines, distincte de l’expérimentation actuelle. Afin que le dispositif soit pleinement opérationnel, la durée de l’expérimentation et les délais de candidature des collectivités ont été calqués sur ceux qui ont été prévus lors de l’examen de la loi Élan. Cela permettra aux collectivités de disposer d’un temps suffisant pour constituer un dossier de candidature,

Notamment, la méthode du carroyage, qui avait été très défavorable à La Réunion, à la Martinique et à la Guadeloupe, n’a pas été retenue. Cette nouvelle géographie inclut dorénavant 247 QPV ultramarins, contre 218 précédemment. En accord avec Mme Bélim, la commission a supprimé l’article 2 pour tenir compte de cette réforme intervenue après le dépôt de la proposition de loi. Enfin, l’article 3 concerne l’élaboration d’un marquage régions ultrapériphériques (RUP) dérogatoire au marquage CE dans le domaine de la construction,

l’entrée en vigueur partielle du nouveau règlement sur les produits de construction et l’exemption pour les régions ultrapériphériques qu’il contient est également une étape décisive.

la question des normes est aussi et peut être même surtout celle des normes volontaires, qui doivent être partagées par l’ensemble des acteurs, permettant tout particulièrement de veiller à l’assurabilité des bâtiments. Nous savons tous combien la question de l’assurabilité devient complexe dans les outre mer, frappés régulièrement et durement par des phénomènes climatiques de plus en plus intenses. En somme, si l’évolution du droit européen est une avancée très importante, les travaux pour aboutir concrètement sont toujours en cours. C’est la raison pour laquelle la commission a, avec l’accord de Mme Bélim, supprimé l’article 3.

mes chers collègues, ce que je souhaitais dire en introduction de nos débats. Je tiens encore une fois à remercier Audrey Bélim de nos échanges constructifs. Je salue sa disponibilité et son engagement en amont de l’examen de cette proposition de loi. En tant que présidente de la délégation aux outre mer, je me félicite que notre agenda parlementaire mette une fois de plus à l’honneur des problématiques ultramarines. La parole

Monsieur le président, madame la présidente de la commission des affaires économiques, chère Dominique Estrosi Sassone, madame

et indignes est supérieur à 150 000, l’habitat informel et dégradé atteint des niveaux records dans certains de nos territoires et l’offre abordable est insuffisante. Ces constats appellent une action forte. continuer à accélérer pour construire plus de nouveaux logements, réhabiliter les logements anciens, lutter contre l’habitat indigne et proposer de vrais parcours résidentiels comportant des logements très sociaux, des logements sociaux, mais aussi des logements intermédiaires et dans le parc libre.

référentiels construction, compétents dans des zones géographiques précisées par décret, afin de contribuer à la mise en œuvre de l’exemption que j’évoquais, en tenant compte des besoins de la production, ainsi que des spécificités et des contraintes locales.

Trop souvent, nos territoires sont les grands oubliés des politiques nationales de logement, alors même que les difficultés y sont exacerbées du fait de loyers inabordables, d’un accès au foncier limité, de normes de construction inadaptées et d’un habitat insalubre. Ce texte a le mérite de proposer des solutions pragmatiques, adaptées à nos réalités locales. Dans nos collectivités ultramarines, notamment à Saint Martin, le logement constitue un enjeu crucial. Les loyers élevés, le manque d’infrastructures adaptées et les difficultés d’accès au logement pèsent lourdement sur nos populations.

Si Saint Martin n’est pas incluse dans la liste officielle des zones dites tendues, en raison de son statut spécifique régi par l’article 74 de la Constitution, son marché immobilier connaît des tensions comparables à ces territoires. Nous faisons face à un fort déséquilibre entre l’offre et la demande, caractérisée par des loyers élevés et un déficit de logements accessibles, notamment pour les ménages les plus modestes. 1 295 logements sont vacants, soit 8,7 % du parc immobilier.

11 % des logements sont des résidences secondaires. Face à cette tension sur le marché du logement, la collectivité de Saint Martin a engagé des actions concrètes pour structurer une politique efficace et durable.

l’offre de logements adaptés, à encourager la réhabilitation du parc existant, à structurer une politique foncière durable et à faire du logement un levier d’attractivité pour le territoire. Le 13 février 2025, la collectivité de Saint Martin a signé une convention tripartite avec le groupe Action Logement et l’État, afin de renforcer l’offre de logements et d’accompagner les Saint Martinois. Ce partenariat structurant permettra de sécuriser les bailleurs, grâce à la garantie locative faciliter l’accession à la propriété, des prêts adaptés, de développer des logements sociaux et abordables, avec Sikoa, et de soutenir les salariés et les entreprises, grâce à des aides ciblées. La mise en œuvre de ce dispositif commencera rapidement. Il constitue une avancée concrète et immédiate pour le logement. Notre priorité est aujourd’hui de stabiliser ces dispositifs et d’accompagner leur mise en œuvre. Ajouter de nouvelles régulations risquerait de complexifier un cadre que nous venons tout juste d’organiser, alors même que nous avons besoin de clarté et d’efficacité. L’adaptation des normes de reconstruction est un enjeu déterminant pour accélérer la reconstruction et garantir des logements durables et accessibles. Grâce au vote intervenu au Parlement européen le 10 avril 2024, notre collectivité pourra désormais déroger au marquage CE pour les matériaux de reconstruction, ce qui constitue une avancée majeure pour notre territoire encore marqué par les séquelles

qui pourraient jouer un rôle essentiel dans l’identification des matériaux adaptés aux réalités locales, en s’appuyant sur l’expertise du bassin caribéen la sécurisation des choix techniques, en impliquant les professionnels du BTP, les scientifiques et les services de l’État, enfin dans la mutualisation des expertises entre les territoires ultramarins, pour éviter la dispersion des efforts et gagner en efficacité. Il est essentiel que cette adaptation se fasse dans un cadre rigoureux et concerté, en lien avec les acteurs économiques et les collectivités concernées. Saint Martin doit être un acteur majeur de cette évolution et tirer parti de cette opportunité pour développer une filière de construction plus autonome, plus durable,

auparavant classé en quartier de veille active, appelait depuis longtemps un accompagnement renforcé. Depuis 2015, les contrats de ville ont permis d’investir plusieurs millions d’euros pour soutenir plus d’une centaine d’actions dans les quartiers prioritaires de Saint

puissent se mettre en place sans obstacle financier. Il nous faut pour cela assurer un financement stable et immédiat pour les politiques de la ville en outre mer. La récente actualisation de la géographie prioritaire a permis d’augmenter le nombre de quartiers concernés, mais elle ne doit pas conduire à un vide budgétaire en attendant la signature des nouveaux contrats.

Monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, nous ne pouvons plus nous contenter de constats. Nous devons agir de façon pragmatique, avec efficacité et en tenant compte des réalités locales. Le logement est un enjeu fondamental pour le développement de nos territoires et pour la qualité de vie de nos concitoyens. Il est donc de notre responsabilité collective d’apporter des réponses durables et adaptées aux défis qui nous font face. À titre personnel, je soutiens pleinement cette proposition de loi, car elle ouvre la voie à des avancées nécessaires pour le logement en outre mer.

ce texte, proposé par notre collègue élue de La Réunion Audrey Bélim, que je salue, vise à répondre aux spécificités des territoires ultramarins en matière de logement. Ces territoires sont en effet marqués par une pression immobilière croissante et des coûts de logement particulièrement élevés, atteignant les niveaux constatés dans les plus grandes villes de l’Hexagone. Nos concitoyens ultramarins doivent également faire face à une offre souvent insuffisante ou peu adaptée aux réalités locales. La rareté du foncier outre mer entraîne des conflits d’usage entre urbanisation, activité agricole et conservation des espaces naturels. Le manque de logements dans les territoires ultramarins est criant. Dans son trentième rapport sur l’état du mal logement en France, tout juste publié, la Fondation Abbé Pierre, nouvellement nommée Fondation pour les logements des défavorisés,

Introduit par la loi Élan du 23 novembre 2018, ce dispositif vise à réguler les hausses excessives de loyer dans les zones dites tendues, où la demande locative est supérieure à l’offre disponible.

Le logement et l’habitat outre mer sont un sujet complexe, qui ne peut pas être réglé en deux heures dans le cadre d’une niche parlementaire, en survolant les sujets. Nous espérons qu’un texte plus complet,

et des normes dans nos territoires ultramarins. Je souhaite notamment alerter sur un point : en l’absence de garantie de la part de l’ensemble des assureurs présents dans nos territoires, la portée d’un éventuel article 3 serait nulle.

est il nécessaire d’égrener la longue liste des mouvements sociaux qui ont jalonné l’histoire de nos territoires ultramarins au cours des deux dernières décennies ? la grève générale de 2009 en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique, le 20 mars 2017, la Guyane se soulève de nouveau. En 2018, Mayotte se déclare « île morte » et les « gilets jaunes » embrasent l’île de La Réunion. De novembre 2021 à mars 2022, les Antilles françaises sont de nouveau le théâtre de violences. Enfin, à l’automne dernier, la Martinique crie son désespoir. Depuis trop longtemps,

Il est plus qu’urgent de remédier efficacement aux inégalités territoriales criantes qui pénalisent les habitants de l’outre mer. Au premier rang de ces inégalités figure l’accès au logement, premier poste de dépenses contraint des Français. En Guadeloupe, les loyers sont aujourd’hui sensiblement les mêmes qu’à Marseille ou à Saint Raphaël. En Martinique, ils sont au niveau du marché locatif bordelais ou lillois. À Saint Pierre et Miquelon, entre mars 2012 et septembre 2023, ils ont progressé de 28,4 %, contre une hausse de 9,1 % au cours de la même période dans l’Hexagone. Ce phénomène s’explique par un déficit de 110 000 logements, alors même que 80 % des habitants sont éligibles au logement social. social. Dans ce contexte de très forte tension – 38 communes ultramarines sont reconnues comme zones tendues – la possibilité d’un encadrement des loyers constituerait un premier outil de régulation du marché et un levier de sanction envers les propriétaires pratiquant des loyers excessifs. Cela offrirait aux classes populaires et aux classes moyennes une plus grande mobilité résidentielle, malgré le défaut d’offre de logements.

nous regrettons la suppression de l’article 3 portant la création de centres scientifiques et techniques du bâtiment des territoires ultramarins. Cette approche prometteuse est considérée comme aboutie par le Gouvernement – M. le ministre d’État l’a indiqué –, ainsi que par les acteurs économiques.

Enfin, pour apporter des réponses durables, cette réforme des marchés du logement ultramarin ne pourra se dispenser ni d’un combat pour des logements décents ni d’une réforme de la gestion foncière, dans un contexte de changement climatique et de transition écologique. Afin de restaurer la qualité du lien entre la République et tous ces territoires, il est urgent que le Gouvernement, en association avec le Parlement,

nous abordons aujourd’hui une thématique importante. La crise du logement qui affecte les outre mer est bien connue. Nous savons tous à quel point la situation est critique, et, comme toujours, le véritable défi est d’apporter des réponses concrètes et efficaces.

? Quels enseignements pouvons nous collectivement retenir des deux plans logements outre mer mis en œuvre depuis 2015 ? Le groupe Union Centriste soutiendra le texte issu des travaux de la commission des affaires économiques.

métropole. Elle laisse toutefois la porte ouverte à d’autres mesures qui, dans bien des cas, sont aussi pertinentes en métropole qu’outre mer. La crise du logement ne doit pas être uniquement abordée au prisme des loyers. Elle appelle un éventail de solutions bien plus large. Qu’il s’agisse de libérer du foncier, de lutter contre la vacance, d’accélérer la rénovation et la réhabilitation ou d’adapter les techniques de construction des bâtiments selon les risques météorologiques locaux, il est évident que nous ne devons pas nous arrêter à une seule mesure. seule mesure. En supprimant l’article 3, qui prévoyait la création de centres d’agrément afin d’homologuer les matériaux de construction dans les territoires ultramarins, de garantir leur qualité et d’établir des référentiels normatifs adaptés aux spécificités ultramarines, la commission a ouvert un débat plus large sur l’impérieuse question de l’adaptation des normes. Il est urgent d’élargir la réflexion, au delà de la construction et de l’urbanisme, à d’autres secteurs clés que sont l’agroalimentaire, la gestion des déchets, l’énergie, l’adaptation au changement climatique, dont les

Que penser de ces calculs au regard de la situation de Mayotte aujourd’hui ? La méthode de carroyage utilisée dans l’Hexagone ne peut pas s’appliquer partout. Le lien humain est une nécessité pour comprendre le territoire et les attentes des habitants. Nous connaissons l’importance de la variable du logement dans les derniers scrutins aux États Unis, en Irlande ou encore en Espagne, et bientôt au Canada. Lorsque les loyers augmentent plus vite que les revenus, entraînant un fossé générationnel dans l’accès au logement, avec des répercussions sur la santé, lorsque les logements sont indécents, tous les ingrédients d’un cocktail explosif Face à ces enjeux, le groupe Union Centriste soutiendra cette proposition de loi et sera au rendez vous des futurs débats sur le logement, en outre mer comme en métropole. La parole

C’est particulièrement vrai en outre mer, où le décalage entre les salaires et le coût de la vie aggrave encore les difficultés et la précarité. Selon les estimations du ministère du logement, les ménages ultramarins doivent faire face à des loyers aussi élevés qu’à Bordeaux, Lyon ou Marseille, malgré une offre limitée et des logements souvent vétustes. Cette situation, à laquelle s’ajoute un taux de pauvreté plus élevé qu’en Hexagone, rend l’accès au logement particulièrement ardu pour les populations les plus précaires.

où le coût des loyers est en décalage avec les besoins. Cet encadrement devrait nous permettre d’endiguer la hausse du prix des loyers, même si nous avons par ailleurs besoin d’une politique de rénovation et de construction de logements sociaux, que l’État refuse de financer depuis bientôt dix ans. Ce n’est pas seulement une question de loyers qui nous est posée ce soir : c’est aussi une question d’habitat et de qualité des logements, au moment où les catastrophes climatiques nous renvoient à l’urgence écologique, que les politiques gouvernementales ont encore trop de mal à appréhender. Il est indispensable de tenir compte des conditions météorologiques particulières dans lesquelles vivent nos compatriotes des outre mer, à qui nous rendons la tâche difficile depuis Paris lorsque nous leur imposons des normes en complète dissonance avec la réalité.

la réalité du climat et à l’isolation thermique des bâtiments. Cette dernière doit être adaptée pour faciliter les constructions et améliorer les conditions de vie de toutes et de tous. Ce qui est certain, c’est que les personnes les mieux placées pour définir et approuver les normes de construction les plus pertinentes sont les acteurs du logement, du bâtiment, les scientifiques, toutes celles et tous ceux qui vivent dans les départements et les régions d’outre mer, qui connaissent leur territoire et ses besoins.

mer. Avec plus de 2,6 millions de demandes de logement social non satisfaites, la crise du logement atteint un niveau alarmant en France. Derrière ce chiffre, ce sont des millions de nos concitoyens qui vivent dans des conditions indignes, peinant à offrir à leurs enfants un foyer stable, propice à leur épanouissement et à leur réussite scolaire. Comme le souligne avec justesse la Fondation Abbé Pierre, « le mal logement est une blessure sociale qui ronge notre pacte républicain ». Cette blessure est d’autant plus profonde dans nos territoires d’outre mer que la fracture économique et sociale avec la métropole ne cesse de se creuser. Aujourd’hui, 75 % des ménages ultramarins éligibles au logement social en sont exclus. Cette réalité heurte autant qu’elle interroge. Car un logement, ce n’est pas seulement quatre murs et un toit : c’est le socle d’une vie digne, la possibilité d’offrir à ses enfants un environnement stable où ils peuvent grandir, étudier et se construire un avenir. Combien d’élèves rongés par la précarité de leur logement peinent à se concentrer à l’école ? Combien de familles s’entassent dans des espaces insalubres, exposées à l’humidité, aux moisissures, à des infrastructures menaçant de s’effondrer ? ? Pour ceux qui ont un toit, la précarité persiste. À Mayotte, déjà bien avant que le cyclone Chido ne frappe, combien de familles survivaient dans des bidonvilles insalubres, sans perspective d’en sortir ? Comment accepter que, en France, en 2025, l’accès à un logement digne soit un luxe inaccessible pour tant de nos compatriotes ? Cette situation est d’autant plus intolérable pour les personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie, qui sont confrontées à un véritable parcours du combattant au vu de la rareté des logements adaptés. Le problème de fond est connu : le coût du logement est devenu insoutenable. En outre mer, les loyers atteignent des niveaux comparables à ceux de la métropole, alors même que 18 % des Français vivant dans la grande pauvreté résident dans ces territoires. Les salaires y sont moins élevés, mais les ménages doivent payer plus. Cette inégalité, nourrie par la spéculation foncière, est inacceptable. Le logement ne peut être traité comme un simple produit de marché. Il est avant tout un droit fondamental. Face à cette crise, nous avons des solutions. des solutions. L’encadrement des loyers, déjà expérimenté avec succès en métropole, doit être institué de manière pérenne en outre mer. Pourquoi ce qui fonctionne ici ne serait il pas appliqué là bas ? Mais agir sur les loyers ne suffit pas. Nous devons aussi garantir des logements durables,

Madame la ministre, notre République ne peut plus détourner le regard. Trop de mesures prises jusqu’ici n’ont été que des pansements sur une plaie béante, ne permettant jamais de s’attaquer aux causes profondes de la crise. Il est temps d’apporter des réponses fortes, à la hauteur des attentes et de la dignité que nous devons à nos compatriotes ultramarins. Ce texte offre de nouvelles perspectives, mais il nous faudra aller encore plus loin,

je veux tout d’abord associer à mes propos notre collègue Saïd Omar Oili, qui, faute d’avion depuis Mayotte, ne peut pas être parmi nous aujourd’hui. Il aurait souhaité s’exprimer sur cette proposition de loi, qu’il soutient avec Avant son examen en commission, ce texte comportait trois pistes de solutions à la crise du logement qui sévit dans les outre mer plus gravement encore qu’en métropole. Les territoires ultramarins, du fait de leurs multiples spécificités, sont en effet frappés plus durement par des réalités économiques, géographiques et climatiques sans commune mesure avec ce que connaît l’Hexagone. Sans vouloir vous assommer de chiffres, je citerai les plus éloquents en outre mer, 80 % des ménages sont éligibles au logement social, mais seuls 25 % y résident. 70 % de la population ultramarine pourraient même légitimement prétendre au logement très

déficit de constructions, coût des matériaux, problème de foncier et de zonage, etc. Pour tous nos concitoyens, qu’ils soient ou non ultramarins, le logement est aujourd’hui le premier poste de dépenses. Cette situation est d’autant plus prégnante dans les outre mer. proposition de loi, notre collègue Audrey Bélim a pour ambition de traiter le problème avec précision et simplicité. L’article 1, conservé par la commission, autorise l’encadrement des loyers dans les communes ultramarines considérées comme tendues. Compte tenu des éléments que j’ai évoqués précédemment et de la forte concentration de la population ultramarine dans le parc privé, la nécessité de rééquilibrer le marché et de donner des outils de régulation aux élus locaux s’impose. L’encadrement des loyers est un dispositif qui a fait ses preuves, puisqu’il permet de bloquer les loyers abusifs au delà de 20 % d’un loyer de référence fixé en fonction des prix du marché. Malheureusement, la publication du décret du 25 août 2023, qui élargissait la liste des communes tendues, est intervenue

Depuis bientôt un an, l’Union européenne autorise la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint Martin à déroger au marquage CE et à importer des produits de construction issus de leur environnement géographique. C’est un gain de temps et d’argent. Cela relève aussi du bon sens écologique : non seulement les seulement les matériaux ont une empreinte carbone plus faible, mais ils sont aussi plus adaptés aux réalités locales. L’article 3, dans sa rédaction initiale, prévoyait ainsi de mettre en place de nouveaux mécanismes locaux de contrôle et de certification des matériaux et de créer des centres d’agrément pour homologuer les matériaux ultramarins.

de La Réunion. La question du logement dans les outre mer est un enjeu majeur. Dans ces territoires, un grand nombre d’habitations sont précaires ou insalubres, exposant leurs habitants à des conditions de vie indignes. Au delà de ces situations critiques, de nombreux foyers sont également confrontés à de véritables problèmes de confort, tels qu’un vis à vis trop proche, une isolation insuffisante ou des niveaux préoccupants d’humidité. En Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et dans bien d’autres territoires encore, l’accès à un logement décent est un véritable défi, et la question de l’accès à l’eau courante en est un exemple frappant. Si la situation de Mayotte a été largement évoquée après le passage du cyclone Chido, d’autres territoires font également face à des coupures d’eau prolongées, qui perturbent profondément le quotidien des habitants et affectent aussi bien les foyers que les établissements publics, tels que les écoles et les hôpitaux. Ces difficultés sont d’autant plus dommageables que les revenus y sont bien inférieurs à ceux de l’Hexagone, tandis que le taux de pauvreté y demeure très élevé. Alors que dans l’Hexagone, une fraction relativement réduite de la population est confrontée à une extrême précarité, la situation dans les outre mer est bien plus préoccupante, notamment aux Antilles et en Guyane, où une large partie des habitants vit en situation de grande vulnérabilité économique. Par ailleurs, à la problématique de la qualité des logements s’ajoute la question de leur insuffisance, en particulier s’agissant des logements sociaux. Si 80 % des foyers ultramarins remplissent les critères d’attribution d’un logement social, seuls 15 % d’entre eux en disposent effectivement. En Guadeloupe, plus de 10 000 demandes de logement social seraient en attente ; il y en aurait 12 000 en Guyane et 45 000 à La Réunion. Face à cette pénurie, des milliers de demandes restent en attente dans chaque territoire, forçant de nombreux habitants à se tourner vers le parc privé. Or les loyers y sont souvent bien plus élevés que dans l’Hexagone. Ils atteignent dans certains cas des niveaux comparables à ceux des grandes métropoles françaises. Mahault, en Guadeloupe, le prix du mètre carré en location dépasse ainsi celui de certaines grandes villes de l’Hexagone, ce qui rend l’accès au logement particulièrement difficile pour les ménages les plus modestes. conséquence directe le poids considérable du logement dans le budget des familles ultramarines. Dans certaines communes de La Réunion, les dépenses liées au logement peuvent représenter 80 % des revenus. Pourtant, lorsque la loi Élan a institué un encadrement expérimental des loyers dans les zones tendues, les territoires ultramarins ont été exclus de cette mesure. Depuis six ans, malgré les revendications constantes des élus locaux, cette expérimentation n’a jamais été étendue aux départements et régions d’outre mer, alors même que la situation y est particulièrement critique.

est précisément l’objet de cette proposition de loi : créer une expérimentation spécifique en matière d’encadrement des loyers dans les Drom, pour une durée de cinq ans. Cette mesure permettra aux collectivités ultramarines qui le souhaitent d’y adhérer librement pendant une période de deux ans. Dans l’Hexagone, près de soixante dix communes appliquent déjà l’encadrement des loyers. Il serait donc profondément injuste de ne pas accorder la même possibilité aux collectivités ultramarines qui en formulent la demande. Cette disposition s’inscrit pleinement dans le combat plus large mené contre la vie chère en outre mer, qui exige des solutions multiples et adaptées aux réalités locales.

Pourtant, depuis son entrée en vigueur, cette mesure convainc partout où elle est mise en œuvre. Ce n’est certes pas une solution miracle ; il s’agit plutôt d’un dispositif de bon sens, qui permet aux élus locaux de tenir les marchés lorsque les prix s’envolent.

Il est prévu que l’expérimentation prenne fin en novembre 2026. À ce jour, le dispositif s’applique dans 69 communes et a vocation à s’étendre, à s’éteindre… La proposition de loi dont nous débattons en est la preuve : les départements et régions d’outre mer pourront bientôt mettre en application cet encadrement des loyers et, ainsi, faciliter l’accès au logement de nombreux ménages ou, au moins, éviter que leurs difficultés ne s’accroissent. Avec ce texte, la crise du logement est aujourd’hui à notre ordre du jour au travers de la situation particulièrement préoccupante des outre mer. Nous ne savons pas quand nous aurons l’occasion de parler de nouveau du droit au logement, lequel ne semble pas être une priorité du Premier ministre.

L’expérimentation actuelle de l’encadrement des loyers arrivera à échéance en 2026. Elle est en cours d’évaluation par le Gouvernement. Or il n’est pas souhaitable de la pérenniser avant de disposer d’un bilan global.

essentiel de disposer d’un bilan de cette expérimentation, afin d’avoir une meilleure compréhension des effets de cette mesure sur le marché locatif, notamment de ses effets de bord éventuels, préalablement à toute décision de pérennisation du dispositif. Ce bilan fera l’objet

pour les conditions d’application d’un complément de loyer, aux règles de décence spécifiques à nos territoires, actuellement fixées par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit déjà un calendrier propre

ma chère collègue, de ne pas appliquer les règles relatives au diagnostic de performance énergétique de l’Hexagone pour cette expérimentation dans les outre mer. Mais je sais également que les règles de décence

au nom de quel principe cela devrait il être autorisé dans les outre mer ? De même, la fourniture d’eau chaude n’est pas obligatoire pour qu’un logement soit considéré comme décent dans les outre mer. Cela se justifie au titre des spécificités ultramarines. Pour autant, autant, un logement sans eau chaude doit il pouvoir faire l’objet d’un complément de loyer, même dans les outre mer ? Même s’ils sont considérés comme décents, quelque 22 000 logements sont jugés comme précaires à La Réunion et 9 % du parc de logements ne disposent pas d’eau chaude sanitaire. C’est ce que je mettais en évidence en 2022 avec Victorin Lurel et Guillaume Gontard dans notre rapport sur la politique du logement dans les

Il s’agit de critères qui avaient été initialement pensés pour le territoire hexagonal, le seul concerné jusqu’à présent par l’expérimentation, et qui sont manifestement inadaptés aux territoires d’outre mer. les critères actuellement prévus par la loi Élan, on trouve les signes d’humidité sur certains murs, des fenêtres qui laissent anormalement passer l’air, hors grille de ventilation, ou encore une mauvaise exposition de la pièce principale. sans le présent amendement, en outre mer, toute construction qui présenterait des signes d’humidité sur certains murs, ce qui est fréquent compte tenu des conditions climatiques locales, ou qui disposerait d’un dispositif de ventilation naturelle, ce qui est de bonne pratique, ne pourrait paradoxalement

Le présent amendement vise, à juste titre, à adapter à l’outre mer les critères de déclenchement du complément de loyer, en renvoyant aux critères généraux de décence prévus par la loi du 6 Il s’agit notamment de l’absence de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, de l’absence de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites et d’un niveau de performance énergétique adapté à l’outre mer.

En outre, toute modification des critères de délimitation de la géographie prioritaire de la ville nécessite un calibrage fin. Les critères de délimitation des QPV dans les outre mer sont spécifiques à ces territoires et ne se superposent pas à ceux qui sont utilisés dans l’Hexagone. l’Hexagone. La rédaction actuelle de la loi Lamy, n’induit donc pas un accès plus restrictif des territoires ultramarins à la politique de la ville : avis défavorable.

la mission sera d’appliquer l’exemption de marquage CE, de soutenir l’innovation locale et de définir des référentiels de construction adaptés à nos spécificités et aux besoins de la production locale. Ces comités devront intégrer en leur représentants des filières de construction, scientifiques, experts… –, garants de leur pertinence et de leur efficacité. La rédaction que je vous propose procède d’une concertation avec les cabinets de Manuel Valls et de Valérie Létard, France Assureurs, l’Agence Qualité Construction et la Fédération des entreprises d’outre mer. En outre, elle est soutenue par le Bureau de normalisation des techniques et équipements de la construction du bâtiment et par le Conseil national de l’ordre des architectes. À l’issue de longs échanges, nous avons abouti à une rédaction faisant consensus, preuve que toutes les parties sont prêtes à avancer sur le sujet. L’adaptation des normes n’est plus une option, c’est une nécessité. Quel est l’avis de la

pour faire enfin aboutir les initiatives visant à adapter les normes, en nous appuyant sur les évolutions récentes du droit européen.

Madame la ministre,

Merci